demande du groupe Les Républicains, de la proposition de résolution visant à affirmer la nécessité d'un accord ambitieux lors de la COP26 de Glasgow permettant de garantir l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « Il est temps de dire : " Assez ! " Assez de brutaliser la biodiversité ; assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone ; assez de traiter la nature comme des toilettes ; assez de brûler, forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes. Ces mots ont été prononcés par António Guterres, secrétaire général de l'ONU, à Glasgow, pour l'ouverture de la COP26, il y a quelques heures. Près de cinquante ans après le premier Sommet de la Terre, à Stockholm, ces mots ont une résonance particulière : ils traduisent l'urgence climatique. cinquante ans, depuis cette première prise de conscience, notre environnement et la biodiversité terrestre n'ont cessé de se détériorer. Entre 1970 et 2016, près de 68 % des populations de vertébrés ont disparu.

Depuis cinquante ans, le nombre de catastrophes climatiques a été multiplié par cinq. Il ne passe pas un jour sans que l'actualité nous donne à voir des images d'inondations, de sécheresses, de tempêtes dévastatrices. Il n'existe pas un seul élu local qui ne soit pas inquiet des conséquences du dérèglement climatique pour sa commune et ses concitoyens. Pendant longtemps, le réchauffement climatique n'apparaissait pas comme une réalité immédiate aux yeux de beaucoup et parler de l'impact de nos industries et de notre consommation sur l'environnement était presque un tabou. Il aura finalement fallu attendre le 12 décembre 2015, c'est-à-dire la vingt pour qu'un accord soit adopté sous le nom d'accord de Paris. Cet accord historique engage les signataires à poursuivre leurs efforts pour limiter l'augmentation de la température de 1,5 degré Celsius et avec pour objectif une limitation de la hausse de la température moyenne de la planète à moins de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels. Alors que les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, la possibilité de parvenir à un accord international contraignant et à un engagement fort des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre semble toujours aussi complexe. C'est tout naturellement que le groupe de travail Enjeux internationaux-climat-environnement-développement, sous l'impulsion de son président Ronan Dantec,

Cette résolution, nous l'avons déposée afin de rappeler la responsabilité de la France sur ce sujet et de réaffirmer aussi le rôle de notre pays comme moteur dans les négociations internationales. L'accord de Paris nous engage particulièrement, parce qu'il a été signé sur notre sol, et nous devons garantir sa mise en oeuvre effective. Avec la volonté, l'engagement et le soutien du président Gérard Larcher, le Sénat a su se mobiliser depuis plusieurs années pour réfléchir, débattre et proposer des solutions concrètes pour prévenir et lutter contre les effets du dérèglement climatique. Cette réflexion, nous l'avons menée afin de donner aux élus locaux, de plus en plus préoccupés par les risques de catastrophe naturelle, les moyens d'agir et de décliner dans les territoires des politiques innovantes. La France a une double responsabilité dans ces négociations

Avec pragmatisme et détermination, en constatant les effets du dérèglement climatique dans nos territoires, nous avons entamé une réforme profonde de nos modes de consommation et de production afin de diminuer l'impact de l'homme sur l'environnement, de préserver notre biodiversité et nos paysages. En 1995, la France adoptait la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui inscrira dans le code de l'environnement que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation Le Grenelle de l'environnement a également marqué un tournant qui a engagé progressivement notre pays et nos concitoyens vers une transition profonde de nos modèles de consommation et de production, vers un modèle qui parvient à concilier avec succès économie et écologie. Mes chers collègues, la transition verte n'a jamais été synonyme de décroissance ; elle est avant tout une chance formidable de création d'emplois et d'innovations. Hydrogène vert, décarbonation de notre industrie, innovation sur le nucléaire, moyens de transport décarbonés, véhicule électrique, etc. : les entreprises françaises sont d'ores et déjà mobilisées sur tous ces chantiers et nous avons le potentiel pour en assurer le leadership. Notre pays est désormais en mesure de montrer l'exemple sur la scène internationale, de montrer qu'il est possible de concilier croissance et décarbonation. Bien évidemment, je comprends les associations et les citoyens qui voudraient aller plus vite et plus loin. Devant l'urgence, on pourrait volontiers leur donner raison et satisfaction ; néanmoins, pour que la transition verte soit acceptable et acceptée par chacun de nos concitoyens, Le tri sélectif, la lutte contre le gaspillage, la modalité, la rénovation des bâtiments, l'achat en circuit court, etc. : nos concitoyens sont les premiers acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique. Les collectivités locales, les institutions et l'État sont engagés, leur rôle est essentiel pour l'exemplarité, bien sûr, et pour l'impact positif de leurs actions. Le changement s'impose désormais en profondeur et au quotidien. Ce serait un mauvais signal que celui qui consisterait à imposer un changement radical, brutal, en quelques semaines ou quelques mois. Il nous faut encore du temps pour développer les innovations, du temps pour mettre en place les bonnes pratiques, du temps pour former les ingénieurs et conforter les métiers de la croissance verte. Et il n'y a là rien de contradictoire avec l'urgence que j'évoquais au début de mon propos : il faut laisser du temps à chacun. Bien entendu, l'engagement français n'est pas seul suffisant et l'enjeu climatique est avant tout un enjeu international. Je ne puis que saluer les engagements de l'Union européenne, moteur dans la lutte contre le dérèglement climatique, qui a notamment fixé des objectifs ambitieux. C'est en tirant parti de cette impulsion, en coopérant avec nos voisins européens, que nous parviendrons véritablement à réduire nos émissions et à peser sur les pays plus émetteurs que nous. Le paquet Climat présenté en juillet dernier prévoit des mesures d'une ampleur inédite, notamment la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, l'extension et le renforcement du marché européen du carbone ou encore la fin de voitures thermiques pour 2035. Le « vieux monde »- c'est ainsi que l'on appelait l'Europe -est en pleine renaissance. Dans quelques jours, nous pourrons évaluer le bilan de la COP26 de Glasgow sera-t-elle un échec, comme le prédisent certains, ou plutôt une réussite, comme je le souhaite ardemment, avec beaucoup d'entre nous ? Un succès constituerait un formidable message d'espoir pour la planète ; j'irai jusqu'à dire que cela serait une véritable espérance pour la jeunesse, qui aspire à vivre dans un monde où l'horizon s'éclaircirait enfin. C'est cette petite flamme qu'il nous appartient de préserver et de transmettre pour la faire grandir. La parole est

Il est vrai que la négociation internationale sur le climat nous a habitués à tant de discours définitifs, la main sur le coeur, sur la nécessité d'agir à la hauteur de ce défi absolu pour l'avenir de l'humanité que toute nouvelle déclaration ou résolution, tout nouvel engagement sont évidemment sujets à caution, suscitent scepticisme, voire ironie, tant ils ont été généralement peu suivis par les actes qu'ils claironnaient. Je ne l'ignore pas ; néanmoins, je suis fier de pouvoir vous présenter avec mes collègues Didier Mandelli et Jean-François Longeot cette proposition de résolution, nourrie des auditions et des remarques du groupe de travail Enjeux internationaux-climat-environnement-développement, que j'ai l'honneur de présider. Une proposition de résolution de ce type envoie déjà un premier message important : le soutien que la représentation nationale apporte aux négociateurs français et européens en leur demandant de rester les moteurs de la négociation climatique internationale, de préserver la dynamique de l'accord de Paris, accord complexe et probablement incomplet, mais qui reste à ce stade le seul socle de négociation multilatérale sur le climat. Ce message pourra aussi être délivré dans les autres instances et lieux internationaux où interviennent les sénatrices et sénateurs français, notamment l'Union interparlementaire (UIP) ou l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), voire, plus largement, dans le cadre des groupes interparlementaires d'amitié. Cette proposition de résolution ne se limite justement pas à un simple souhait d'accord ambitieux à Glasgow, mais dessine aussi des pistes pour un monde de stabilité climatique. Nous le disons dans plusieurs paragraphes : sans intégration des enjeux de développement, nous ne pouvons espérer construire les nouvelles régulations dont nous avons besoin. Ainsi, nous rappelons le caractère impératif de l'atteinte de l'enveloppe annuelle de 100 milliards de dollars pour les pays les moins développés, engagement que les pays riches avaient pris à Copenhague, il y a déjà douze ans. De manière plus prospective- et nous avons fait ici le choix d'une proposition de résolution qui entre un peu dans la complexité et la technicité de l'accord de Paris -, nous insistons sur l'importance d'une mobilisation prioritaire des futurs fonds de compensation vers les pays en développement, en particulier ceux du continent africain.

aux pays en développement de participer à l'effort de stabilisation du climat, d'être finalement solidaires des pays émetteurs historiques, si, dans le même temps, nous ne leur accordons pas un accès garanti en nombre suffisant aux vaccins contre le covid-19. Le monde de l'accord de Paris est un monde toujours un peu utopique, un monde où la communauté des États a compris que ses intérêts vitaux étaient plus dans la coopération que dans l'affrontement- logique, qui ne s'impose malheureusement que très rarement de manière le tragique de l'Histoire nous le rappelle. Les inventeurs de l'architecture de cet accord de Paris étaient évidemment conscients de cette difficulté, du caractère finalement un peu contre nature de ce pari sur l'intelligence collective des États à dépasser leurs intérêts immédiats pour leur avenir commun. Aussi, ils ont proposé des mécanismes de coopération plus opérationnels entre États volontaires : c'est le sens de l'article 6, dont la finalisation a déjà bloqué deux COP et dont nous soulignons l'importance. Ce n'est pas sans raison. Derrière cet article, c'est potentiellement une nouvelle géographie économique du monde qui se dessine. D'un côté, de nouveaux espaces de coopérations où se transfèrent des tonnes de CO2 entre États partageant des objectifs communs de réduction des émissions, une nouvelle guerre économique entre grands blocs économiques régionaux n'estimant pas devoir développer les mêmes efforts et dressant entre eux des taxations carbone à leurs frontières. En s'intéressant à ces articles 6 et 13, notre proposition de résolution fait aussi, me semble-t-il, oeuvre de pédagogie en rappelant que la négociation climatique n'est pas seulement une négociation environnementale, mais qu'elle est un des lieux- si ce n'est le premier lieu -où s'écrivent les grands équilibres économiques et géopolitiques de demain. Enfin, en écho à la résolution de notre ancien collègue Jérôme Bignon, adoptée voilà déjà six ans, nous rappelons le rôle essentiel de l'action territoriale, l'importance des politiques engagées par les collectivités pour décliner les objectifs de l'accord de Paris. Une part importante des émissions de CO2 est liée à la vie quotidienne, à la manière de se loger, de se nourrir, de se déplacer. Qui mieux que les élus locaux dispose de cette capacité à agir ? Porte-parole de réseaux de collectivités territoriales internationales dans les négociations climatiques depuis une douzaine d'années, je connais la difficulté que rencontrent les collectivités territoriales à être totalement associées, alors que, pourtant, bien des contributions déterminées au gagneraient en ambition si elles intégraient le potentiel d'action de leurs gouvernements locaux. La France, porteuse au moment de la COP21 de l'agenda de l'action,

les tensions géopolitiques, les conflits et les tentations de repli qui les accompagnent, il y a des idées, chères à notre pays, dont l'importance doit être plus que jamais rappelée : la foi dans l'universel et le multilatéralisme. Car nous ne résoudrons pas une des plus graves crises traversées par l'humanité- le réchauffement climatique et l'extinction de masse de la biodiversité -sans coopération et régulation internationales. En 2015, au Bourget, c'est cette conviction qui avait guidé notre diplomatie et qui avait permis la conclusion du premier accord universel sur le climat, l'accord de Paris. Six ans après, les États signataires se retrouvent à Glasgow pour une COP26 lourde d'enjeux. Formons le voeu que l'universel et le multilatéralisme prévalent de nouveau pour défendre l'acquis de Paris, unique cadre juridique à même de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète à un niveau acceptable pour notre espèce. Nous le savons, cela n'est pas gagné : plusieurs États n'ont toujours pas soumis leur feuille de route aux Nations unies, comme le prévoyait pourtant l'accord de Paris. Pis, peut-être, la somme des engagements aujourd'hui déposés ne permettrait de contenir l'élévation des températures qu'à 2,7 degrés centigrades, niveau qu'on peut juger dramatique à la lecture du récent rapport du Groupe Malgré tout, au grand dam de ses contempteurs, l'accord de Paris fonctionne. Les faits le démontrent : beaucoup d'États jouent aujourd'hui le jeu et respectent le mécanisme créé par la COP21 en soumettant de nouvelles contributions déterminées au niveau national plus ambitieuses que les précédentes. Même la Chine, méfiante à l'égard du multilatéralisme, a déposé sa contribution la semaine passée. Cela étant dit, tout, pour ainsi dire, reste à faire, pour garantir que ces engagements ne soient pas de simples coquilles vides. Ce sera l'un des grands enjeux de la COP26, comme nous l'avons rappelé dans la proposition de résolution qui vous est présentée aujourd'hui. présentée aujourd'hui. Il importe, d'une part, qu'un mécanisme de transparence robuste soit enfin établi en application de l'article 13 de l'accord : ce mécanisme sera le garant de la réciprocité de l'action climatique et de la bonne foi de chacun à s'engager sur la trajectoire de la neutralité carbone. Il convient, d'autre part, d'arrêter enfin les règles du mécanisme du marché du carbone prévu à l'article 6, qui contribueront à donner un signal prix mondial en faveur de la décarbonation et à financer les actions d'atténuation menées par les États les plus vertueux. Pour embarquer l'ensemble des États de la planète dans l'effort climatique, nous devons par ailleurs tenir nos promesses, en mobilisant, comme prévu en 2009, 100 milliards de dollars de financements pour le climat en faveur des pays du Sud. La France respecte ses engagements en la matière. Ce n'est pas le cas de tous les pays. La mobilisation de ces fonds est impérative. Sans elle, il est illusoire d'espérer que les pays en développement, particulièrement ceux du continent africain, prennent avec nous le chemin de la neutralité carbone. Voici quelques-uns des messages que nous avons souhaité adresser au moyen de cette proposition de résolution. La délégation de notre commission, qui représentera le Parlement français à la COP26, portera ces messages dans les échanges qu'elle aura avec nos homologues des autres pays. Elle défendra modestement ces deux idées chères que j'ai évoquées au début de ma prise de parole : l'universel et le multilatéralisme. La parole est à M. Éric Gold.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'accord de Paris obtenu le 12 décembre 2015 constitue un tournant historique des conférences des parties sur le climat en ce que, pour la première fois, les 196 parties se sont engagées à respecter l'objectif de contenir à 1,5 degré Celsius la hausse mondiale des températures d'ici à 2100 par rapport à l'ère préindustrielle. Tel est le défi majeur du XXI siècle qui implique un bouleversement des modes de production, de consommation et de vie de nos sociétés. Après cet état de grâce diplomatique, puis les échecs des COP qui ont suivi, vient le temps d'un premier bilan quinquennal de l'action climatique. Ce travail révèle la nécessité d'accélérer les efforts et d'aboutir à un nouvel accord lors de la COP26 qui se tient en ce moment à Glasgow.

-nous mène vers une trajectoire de 2,7 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle, à condition qu'ils soient effectivement respectés. Or la première partie du sixième rapport d'évaluation du GIEC publié en août dernier souligne qu'une hausse de 2 degrés signifie un dépassement des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture et la santé publique. Certaines conséquences du dérèglement climatique sont jugées « irréversibles pour des siècles ou des millénaires », comme l'acidification des océans, la fonte des glaciers et calottes polaires et l'augmentation du niveau de la mer. Quel que soit le scénario étudié par l'organisme, nous dépasserions la barre de 1,5 degré Celsius dès 2030-2040- à moins d'agir immédiatement et radicalement, ce qui est peu probable. Le secrétaire général des Nations unies a affirmé que cela supposerait sept fois plus d'ambition. Dans le seul secteur de l'énergie, il faudrait renoncer à toute exploitation de l'énergie fossile et atteindre une hausse de 4 % de l'efficacité énergétique par an, soit trois fois plus que pendant les dernières décennies, si l'on s'en tient aux chiffres avancés par l'Agence internationale de l'énergie. Il existe donc un fossé entre le concept et sa réalisation. La proposition de résolution rappelle, à juste titre, que ces engagements doivent être déclinés aux niveaux national et local. En 2020, la crise du covid-19 n'aura finalement eu qu'un impact modeste, moyennant une réduction de 5,4 % des émissions de CO2 dans un monde qui a dû rester à l'arrêt pendant plusieurs mois. C'est cet effort qu'il conviendrait de maintenir de manière annuelle. Est-ce réaliste en l'état actuel des engagements et de leur exécution ? Non. C'est bien la preuve qu'il nous faut à la fois plus d'investissements, plus d'innovation, et surtout plus de sobriété. Le progrès est nécessaire, des technologies de rupture surgiront, mais il n'y aura pas de miracle. Pour ne prendre que les exemples de l'hydrogène ou de la fusion nucléaire, de la capture du CO2 ou encore de la géo-ingénierie, ces innovations et leur diffusion à grande échelle sont essentiellement attendues après 2050. Il sera alors trop tard pour freiner l'emballement du climat. se produira pas davantage de miracle si subsiste une confiance aveugle dans les mécanismes de marché. On pourra imaginer tous les systèmes de compensation carbone possibles pour atteindre la neutralité carbone, d'autres leviers demeurent indispensables réglementation environnementale, investissements massifs publics et privés, taxation du carbone, recherche, formation, etc. Le bilan annuel de l'action climatique du programme des Nations unies pour l'environnement, publié la semaine dernière, déplore des des objectifs de neutralité carbone « vagues, souvent incomplets et non alignés avec la plupart des plans à court terme ». Telle est bien la limite de l'accord de Paris : l'impossibilité de mettre en place un mécanisme de sanctions en cas de non-respect des engagements. La France n'a d'ailleurs pas respecté son premier budget carbone. La COP doit absolument avancer sur les règles de transparence en matière de suivi des réalisations des engagements de chaque État partie. Les conséquences du changement climatique frappent en premier les pays en développement. Il est donc impératif de régler la dette climatique, de convaincre le bloc des responsables historiques de la pollution de respecter enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les accompagner, conformément aux engagements pris à Copenhague en 2009. Au lendemain du G20 qui s'est tenu à Rome, ce dossier ne sera réellement débloqué qu'en 2023, avec trois ans de retard. La prise de conscience s'accroît. Tous les acteurs s'y mettent, avec plus ou moins d'enthousiasme citoyens, entreprises, investisseurs, mais aussi la plupart des États qui ont adopté l'objectif de neutralité carbone selon des échéances allant de 2040 à 2070- à commencer par les pays du G20, responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de serre. L'humanité va devoir s'affranchir des contraintes techniques et financières tout en s'accommodant des limites planétaires pour rendre cet avenir commun encore désirable. Les budgets carbone consommés jusqu'à présent doivent être restitués à ceux qui n'ont pas eu cette chance, à savoir les pays les plus vulnérables, mais aussi aux générations futures. Il revient aux États de gouverner la crise climatique de manière volontariste, coordonnée et juste. Nous voterons la proposition de résolution en espérant sincèrement que la COP26 accouche d'un accord nettement plus ambitieux. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, si je salue l'initiative de cette proposition de résolution, je me permets de saisir l'occasion qui se présente pour dénoncer l'inaction de la France à l'égard de ses engagements climatiques internationaux. Ce texte souligne, à juste titre, le « devoir d'exemplarité des pays moteurs de l'action climatique » dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or l'exemplarité est le dernier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la politique environnementale de la France. Depuis l'accord de Paris, jamais notre pays n'a tenu ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La condamnation historique de l'État dans le cadre de « l'affaire du siècle » et la décision inédite rendue au début du mois de juillet par le Conseil d'État, qui demande au Gouvernement de « prendre toutes mesures utiles permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre », mettent en lumière l'inaction du pouvoir en place. Le Président de la République annonçait en mai 2020 vouloir « changer la nature même de la mondialisation » afin de répondre à l'urgence écologique. Cette volonté se traduit par une distribution massive d'argent public, sans condition, aux secteurs de l'automobile et de l'aviation. Le même président, lors de son discours sur la France de 2030, a fait part de son souhait d'explorer les fonds marins, riches en métaux et hydrocarbures. Cette soudaine envie d'aventure ne traduit rien d'autre que les prémices d'une exploitation de ces espaces. Si le président s'en défend, je demande donc pourquoi la France s'est abstenue lors de l'adoption par l'Union internationale pour la conservation de la nature un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. La solidarité internationale doit jouer un rôle primordial dans l'action climatique. Les pays développés s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an en 2019, le fonds à destination de ces pays n'atteignait que 80 milliards de dollars. La COP de Glasgow doit donc compenser ce retard. Là aussi, la France devrait prendre ses responsabilités. La faible volonté politique de notre exécutif dans la lutte contre le changement climatique nous décrédibilise sur la scène internationale. J'espère que cette proposition de résolution lui permettra d'en prendre davantage conscience. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans mon ultime intervention lors de l'examen de la loi Climat et résilience en juillet dernier, j'invitais le Gouvernement et la majorité sénatoriale à se montrer plus offensifs pour combattre l'insécurité écologique qui sera désormais notre quotidien. Si la France est « sortie des clous » de la trajectoire carbone qu'elle s'était fixée, il n'en demeure pas moins vrai que le quinquennat précédent nous a conféré une légitimité profonde dans la lutte contre le réchauffement climatique, par la signature de l'accord de Paris en 2015. Charge à notre exécutif de mesurer l'héritage de ce leadership écologique édifié sous François Hollande et d'en être à la hauteur dans les négociations internationales qui s'ouvrent en Écosse. C'est donc avec un véritable espoir que je cosigne cette proposition de résolution transpartisane affirmant la nécessité d'un accord ambitieux lors de la COP26 qui commence cette semaine à Glasgow. Certains pourront critiquer, d'autres minimiser ce texte d'appel. Il s'agit néanmoins là d'un geste politique qui honore notre institution en matière environnementale. Parce que mon groupe politique et moi-même sommes convaincus que nous ne pouvons plus, sans cesse, reculer devant l'obstacle, cette résolution se veut, non pas un blanc-seing, mais la traduction minimale de ce que nous attendons des positions défendues à Glasgow par la France- d'autant plus que la tâche ne sera pas facile, le contexte international tendu pouvant grandement nuire à l'accord que la planète attend. On a beaucoup moqué Greta Thunberg en France et ailleurs. Or cette jeune fille, suivie par de nombreux jeunes, a le courage de la raison, tout comme les milliers de scientifiques qui appellent les décideurs à agir d'urgence. Le GIEC confirme les perspectives chaotiques qui sont devant nous : l'enjeu est bien l'extermination ou la survie du vivant.

Si le monde continue sur sa lancée, un réchauffement de 2,7 degrés Celsius est assuré, soit un résultat bien supérieur à 1,5 degré Celsius, et nous condamne à la « catastrophe climatique » selon les mots du secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Aussi, madame la secrétaire d'État, pour sortir des postures de Cassandre, cette résolution vous donne une feuille de route, ou plutôt une feuille de rappel des objectifs que nous nous sommes fixés lors des accords de Paris, afin que la France ne soit pas inactive sur le plan climatique Nous souscrivons d'autant plus à cette résolution qu'elle prend en compte la dimension sociale de ce défi de l'humanité ainsi que la dimension solidaire qui incombe aux pays les plus développés et les plus émetteurs envers les États les plus vulnérables et les plus pauvres. Ce point est essentiel, sachant que nous ne sommes toujours pas arrivés à constituer le fonds de 100 milliards de dollars par an à destination des pays en voie de développement. Ce sujet du financement est d'autant plus pressant que la promesse de ce fonds, faite en 2009 à Copenhague, porte sur les cinq années 2020-2025. Selon les dernières projections de l'OCDE, l'objectif ne pourrait être atteint qu'en 2023 ! Encore une fois, nous sommes loin du compte, comme le concède Alok Sharma, le président de la COP26. La solidarité est bien au coeur du virage écologique et philosophique nécessaire pour contenir le réchauffement. Ainsi, cette proposition de résolution rappelle très justement le « caractère impératif de l'atteinte de l'objectif d'une mobilisation par les pays développés de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 Au-delà de cet échec retentissant de la diplomatie climatique mondiale, le retour en scène des États-Unis peut cependant nous redonner quelque optimisme, rapidement tempéré par l'annonce de l'absence des chefs d'État russe, chinois et turc à la COP26. Cette proposition de résolution formulée par la Haute Assemblée dans une quasi-unanimité est aussi l'occasion de rappeler que la question de la diplomatie climatique est également une question démocratique. Sans adhésion des populations, sans justice sociale, nous ne pourrons effectuer l'effort immense de transformation et d'anticipation nécessaire pour l'atténuation Enfin, comme le rappelle ce texte à la suite de Valérie Masson-Delmotte, les collectivités locales ont un rôle éminent à jouer en la matière, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'influence humaine sur le climat global. C'est aussi une histoire d'aménagement du territoire, qui peut aggraver les effets d'un climat qui change. Le défi est colossal. Il concerne chacun d'entre nous et le monde entier. Les États ont une responsabilité encore jamais éprouvée. Toutefois, rien n'est écrit d'avance et cette semaine sera cruciale pour la planète- en cas d'échec, comme en cas de réussite. Cette proposition de résolution vous invite, madame la secrétaire d'État, au courage des actes

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « Comment pouvons-nous danser quand notre terre tourne, comment dormons-nous, alors que nos lits brûlent ? » Voilà ce qu'écrivait en 1987 celui qui fut ministre de l'environnement en Australie de 2007 à 2010. Je veux parler de Peter Garret, plus connu comme leader du groupe de rock Midnight Oil, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui signa avec la chanson un manifeste que les participants à la COP26 pourraient reprendre à l'unisson. effet, la COP26 donne le coup d'envoi d'une décennie décisive qui sera celle du triomphe ou de la tragédie. Elle doit constituer un test de crédibilité et une échéance clé pour au moins deux enjeux au coeur des négociations multilatérales sur le climat la dynamique d'ambition collective enclenchée par l'accord de Paris et le financement du climat promis lors de la COP15 de Copenhague. Les accords de Paris étaient le temps de la promesse, Glasgow doit être celui de l'engagement. C'est le sens de la résolution qui nous est proposée et qui fait suite au travail mené depuis plusieurs mois par notre assemblée, notamment par le groupe d'études présidé par notre collègue Ronan Dantec, qui a procédé à plusieurs auditions sur un sujet désormais placé tout en haut de la pile

à laquelle les pays doivent soumettre des engagements nouveaux et renforcés à l'horizon 2030 ainsi que des stratégies à long terme de développement de faibles émissions de gaz à effet de serre- généralement à l'horizon 2050. La COP26 marque la première étape du mécanisme d'ambition de l'accord de Paris, et un premier test pour sa crédibilité. Le tableau n'est pas rose : si les trois quarts des pays ont soumis leurs contributions déterminées au niveau national pour l'action climatique, cela ne représente qu'un peu plus de la moitié des émissions mondiales, quelques « poids lourds » ne répondant toujours pas à l'appel.

d'ici 2053. Les efforts remarquables de l'Afrique du Sud qui a déposé une CDN très ambitieuse sont également à noter. Même si des avancées sont possibles au cours de la COP26 sur ces engagements à court terme, le fossé sera loin d'être comblé. Raison de plus pour nous rappeler que l'ambition ne peut être réduite aux seuls chiffres des CDN. Des progrès ont été réalisés aux niveaux national et sectoriel, en matière de gouvernance, d'objectifs et de politiques et la proposition de résolution que nous examinons est clairement tournée dans

qui rappelle que le cadre de l'Union interparlementaire peut constituer un levier efficace pour « faciliter la conduite d'un accord ambitieux à l'échelle internationale et sa déclinaison dans les politiques publiques nationales.

Le deuxième objectif qui jalonne cette COP26 est le financement, et plus précisément la promesse faite par les pays développés lors de la COP15 de Copenhague de 2009 de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 auprès de sources publiques et privées pour répondre aux besoins des pays en développement. Cette promesse n'a pas été tenue, puisque 20 milliards de dollars manquent à l'appel.

pourrait être significativement compromise. De la même manière, la réduction de la consommation de charbon est l'un des principaux domaines dans lesquels de nouveaux engagements sont espérés. Après un été marqué par des catastrophes climatiques à répétition et, dans un cruel parallèle, par la sortie d'un nouveau rapport alarmant du GIEC, de nombreux pays demandent aujourd'hui une augmentation de l'adaptation.

À Glasgow, la France s'appuie sur trois mots clés : confiance, transparence et cohérence. Elle est une bonne élève du financement de la lutte pour le climat, avec 6 milliards d'euros par an ; côté engagement, nous partageons notre bonne marche avec l'Union européenne, avec un objectif de baisse de 55 % des émissions d'ici à 2030 et la neutralité carbone en 2050. Néanmoins, le chantier reste vaste, puisqu'il s'agit désormais de répartir l'effort française du Conseil de l'Union européenne, au premier semestre 2022, sera l'occasion d'avancées significatives sur ce dossier. La réussite de la COP21 et des accords de Paris a suscité un formidable espoir à travers le monde. Depuis lors, malgré des avancées, cet espoir a été déçu. La COP26 de Glasgow doit ranimer la flamme.

Passé le temps de l'euphorie, nous devons nous tourner vers des propositions peut-être moins ambitieuses, mais bien plus réalistes. La communication c'est bien, mais l'engagement concret c'est mieux Notre jeunesse, à la pointe, fait entendre sa voix partout dans le monde. Nous devons l'épauler et nous montrer à la hauteur de ses espérances et des enjeux. du territoire et du développement durable, travaille régulièrement sur la problématique climatique à laquelle nous essayons d'apporter des solutions pragmatiques et efficientes.

Le groupe Les Indépendants défend une écologie libérale, une écologie de progrès et d'efficacité, qui s'attache à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. À nos yeux, la solution réside dans la recherche, dans l'innovation et dans l'investissement dans les technologies d'avenir.

Un mix équilibré est nécessaire, entre énergies renouvelables et nucléaire. Il semble que, s'agissant des premières, si la recherche continue à progresser, l'hydrogène et le solaire tiennent la corde. À ce titre, je renouvelle l'appel fait sur l'inclusion de la filière nucléaire dans la taxonomie verte européenne. Les investissements sont nécessaires dans ce domaine et la finance verte, elle aussi, doit être ancrée dans la réalité. Nous devons faire de la crise que nous traversons une relance efficace qui serait un outil au service des transitions. Nous avons tous la responsabilité, à notre niveau, de faire vivre ces transitions et les collectivités ont un rôle primordial à jouer, ainsi que le rappelle cette proposition

Plus graves encore sont les absences de la Chine et de la Russie, respectivement premier et quatrième plus gros émetteurs mondiaux de CO2. Ces absences ne sont pas seulement dues à la pandémie mondiale que nous vivons : nous connaissons depuis longtemps le grand sens de la solidarité internationale Les enjeux climatiques se retrouvent ainsi prisonniers des tensions géopolitiques, et parfois internes. Cela évoque un serpent qui se mord la queue, alors que l'on entrevoit les tensions internationales que provoqueront- et provoquent déjà -les crises climatiques. Les nuages noirs s'amoncellent dans le ciel de Glasgow. Il nous paraît donc essentiel de permettre aux pays en développement d'accéder à l'énergie et à la neutralité carbone et de les aider dans cette transition. d'un combat commun, mondial : nous serons tous touchés par les conséquences du dérèglement climatique si nous n'agissons pas avec intelligence et pragmatisme. Notre situation géopolitique, politique et économique pourrait être bouleversée de manière irréversible.

On n'arrête pas un peuple qui a faim ! La France et l'Union européenne doivent rester chefs de file, comme le conclut cette proposition de résolution. Je rappelle cependant que, malgré les objectifs que nous avons ouvertement exprimés à travers le pacte Vert européen, nous ne représentons que 10 % des émissions mondiales.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme au moment de la COP21, le Sénat souhaite affirmer la nécessité d'un accord ambitieux pour le climat lors de la COP26. Loin d'un discours évoquant « une COP de la dernière chance » ou « une COP qui ne servirait à rien », cette proposition de résolution transpartisane montre combien l'enjeu du sommet de Glasgow est immense. Le récent rapport du GIEC et les manifestations du changement climatique, de plus en plus nombreuses, doivent pousser l'ensemble des parties prenantes à appliquer et à renforcer l'accord de Paris. Au-delà du nécessaire rehaussement des engagements de chaque État, déjà abordé par mes collègues, je m'attarderai sur deux points essentiels soulevés dans cette proposition de résolution : le décloisonnement entre action climatique et action en faveur de la biodiversité et le soutien à la lutte contre le changement climatique dans les pays en voie de développement. Oui, la communauté internationale, dans son ensemble, s'est emparée de la lutte contre le changement climatique. Les négociations internationales sur la diversité biologique arrivent, quant à elles, timidement sur le devant de la scène, même si la pandémie de coronavirus semble avoir agi comme un révélateur. Le sujet des zoonoses s'est ainsi imposé dans le débat public

Ainsi, climat et biodiversité font l'objet de négociations et d'actions séparées, menées sous l'égide de deux conventions différentes des Nations unies. Pourtant, ces deux sujets sont intimement liés les phénomènes météorologiques extrêmes, les sécheresses, l'acidification des océans entraînent la migration des espèces, des bouleversements des chaînes alimentaires et un appauvrissement en espèces végétales et animales. À l'inverse, l'effondrement du phytoplancton et la déforestation réduisent sensiblement la séquestration du CO2 par ces puits de carbone naturels que sont nos océans et nos forêts. Il s'agit pourtant d'un vrai levier pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette organisation en silos des négociations climatiques est donc dépassée. Il est temps de penser la politique environnementale et les négociations internationales de manière globale, et non secteur par secteur. Les politiques d'atténuation du changement climatique et de maintien de la biodiversité doivent être menées de front.

Cette résolution rappelle également le caractère impératif de la mobilisation par les pays développés de 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en voie de développement, dès 2020. Cet engagement, pris lors de la COP15 à Copenhague, en 2009, n'est à ce jour pas respecté : 80 milliards de dollars ont été mobilisés en 2019, d'après l'OCDE, et le rapport commandé par la présidence britannique de la COP26 estime que la cible ne sera atteinte qu'en 2023. Si la récente feuille de route demandée par la présidence britannique semble indiquer que les financements publics seront à la hauteur dans les années à venir, on peut imaginer que les négociations seront âpres sur le sujet. Plusieurs pistes ont déjà été identifiées. Tout d'abord, l'augmentation des contributions publiques doit se concrétiser. Plusieurs États et de nombreuses banques multilatérales se sont engagés à augmenter leur contribution. La France avait, dès 2015, pris l'engagement de porter la sienne à 5 milliards de dollars par an ; un objectif accompli dès 2019. Nous pouvons nous en féliciter, même si le déséquilibre entre dons et prêts reste trop important. La plus grande incertitude vient cependant des financements privés, qui doivent croître, alors qu'ils étaient en baisse en 2019, selon l'OCDE. La fragilisation des économies que nous venons de connaître ces deux dernières années fait craindre que cette baisse ne se poursuive, mais la mobilisation de tous pour lutter contre le changement climatique est primordiale. L'accroissement des fonds privés est donc capital, car nos institutions publiques ne pourront faire face seules. Madame la secrétaire d'État, comment la France et ses partenaires comptent-ils se mobiliser pour garantir les financements privés vers les pays en voie de développement ? Ensuite, et comme le souligne la proposition de résolution dont nous discutons, une plus grande part de ces fonds doit être affectée à l'adaptation face au changement climatique, dont les manifestations sont de plus en plus importantes. Cette mesure était déjà inscrite dans l'accord de Paris. Pourtant, seulement 25 % des fonds lui ont été consacrés en 2019. Ce soutien est attendu, notamment par les petits États insulaires qui subissent la montée des eaux et qui ont un accès difficile aux financements internationaux. La France doit elle-même revoir l'affectation des sommes qu'elle engage dans cette perspective. Enfin, et surtout, les négociations sur les financements post-2025 doivent faire un véritable bond en avant pour aboutir rapidement. Toujours selon l'OCDE, les pays développés mettraient à disposition 117 milliards de dollars en 2025. C'est un vrai point de départ pour construire une stratégie et une perspective sur dix à vingt-cinq ans, en s'appuyant sur les besoins des pays en voie de développement dans les années à venir, croître sensiblement. Les sujets à traiter lors de cette COP26 sont donc nombreux. Quelques jours seulement après son ouverture, le réalisme nous impose de constater que tous n'aboutiront probablement pas. Le multilatéralisme, en matière de négociations climatiques comme de manière plus large,

pris par l'Inde, qui pourraient inspirer d'autres pays et tendre vers des actions concrètes. Ainsi, ce sommet pourrait tout de même permettre des avancées notables, sur la base du travail accompli en 2015 avec l'accord de Paris. La parole

sa portée n'est que symbolique, mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un symbole. Si aujourd'hui toutes les sensibilités politiques demandent au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la vingt-sixième conférence des parties sur le climat soit une réussite, c'est parce que le moment que nous vivons est grave. Nous avons un pouvoir immense. Nous pouvons soit sauver notre monde, soit condamner l'humanité à un avenir infernal. » Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du secrétaire général des Nations unies. Ils résument parfaitement les 3 949 pages du dernier rapport du GIEC. L'impact de l'homme sur le changement climatique est sans équivoque ; toutes les régions du monde sont concernées ; nous ne sommes plus dans la prévision ou dans la théorie, les effets concrets et dramatiques sont là, partout. Le pourtour méditerranéen est particulièrement affecté, les flammes ont ravagé la Californie et la Sibérie, les eaux ont dévasté l'Europe centrale, le Canada a connu des températures tropicales. plus besoin de graphiques pour mesurer l'impact délétère du dérèglement provoqué par le réchauffement de 1,1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Si le rapport du GIEC dessine des scénarios apocalyptiques, avec un réchauffement pouvant atteindre 5,8 degrés d'ici à la fin du siècle, s'il estime que, en l'état actuel de l'engagement de chaque nation, la trajectoire nous fera atteindre 2,7 degrés durant cette période, il nous propose aussi le chemin de l'espoir, celui qui nous permettrait de maintenir le réchauffement autour de 1,5 degré Croyez-en l'expérience des écologistes que nous sommes : annoncer la catastrophe ne permet que rarement de construire un plaidoyer efficace ! Cassandre n'a pas su empêcher la chute de Troie déclamer la fin prochaine de l'humanité a tendance à tétaniser celle-ci, à l'instar du lapin pris dans les phares d'une voiture. C'est donc sur ce motif d'espoir qu'il nous faut nous concentrer oui, c'est possible, mais il faut faire vite. Le message du GIEC ne souffre d'aucune ambiguïté : il nous reste dix ans pour agir. Chaque jour compte, chaque tonne d'émissions, chaque fraction de degré aura un impact sur notre santé et notre sécurité. Nous n'y parviendrons pas sans respecter nos engagements et sans changer de modèle. Pour contenir le réchauffement autour de 1,5 degré, nous devons baisser nos émissions de CO2 de 45 % par rapport à 2010.

pour permettre à chacun de réviser ses objectifs à la hausse. Pour le moment, l'optimisme n'est pas de mise : les trois principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre n'ont avancé que timidement depuis six ans. La présidence Trump a fait perdre quatre ans aux États-Unis et Joe Biden, malgré des excuses, peine à trouver le chemin de l'action ; la Chine propose la neutralité carbone en 2060 et, à ce jour, son président n'a pas jugé opportun de se rendre à Glasgow l'Inde n'a toujours pas remis sa nouvelle contribution. Que dire de la France, qui est toujours loin des objectifs de 2015 ? Le G20 préalable qui s'est tenu ce week-end n'a pas permis d'avancer,

Dans ce marasme, l'Europe, et particulièrement la France, qui en prendra la présidence en janvier, doit jouer un rôle moteur. Après la loi Climat et résilience qui n'atteint pas ses objectifs, après une condamnation pour inaction climatique, notre pays a fort à faire pour retrouver son leadership. Les discours et les bonnes intentions ne suffisent plus. Emmanuel Macron se rêve en premier de cordée, c'est le moment ou jamais d'indiquer la bonne voie et d'imprimer le rythme. Nous devons repartir de Glasgow avec les nouvelles contributions de toutes les nations, avec les trajectoires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone brandis par les uns et les autres, avec un encadrement strict des marchés du carbone, que nous n'avons pas réussi à mettre en place lors des deux dernières COP, et avec un calendrier commun. Dernier sujet, et non des moindres : nous devons accélérer l'effort de solidarité avec les pays en développement. Nous n'avons pas tenu la promesse faite à Copenhague en 2009 de leur fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 ; nous sommes à peine parvenus à 80 milliards et 70 % de ces montants sont versés sous forme de prêts, aggravant la dette de ces États. Cette aide doit se faire sous forme de dons : en matière climatique, c'est un impératif. Ces financements à destination des pays les plus pauvres ne relèvent pas de notre générosité, mais découlent de notre dette climatique : le G20 est responsable de 80 % des émissions des gaz à effet de serre.

proposition de résolution : il est difficile de comprendre que seuls trois groupes aient été initialement associés à sa rédaction. Lors de la préparation de la COP21, un texte ambitieux avait été construit à la suite de travaux auxquels avaient participé l'ensemble des commissions et des groupes. Il est regrettable que cette procédure n'ait pas été réitérée.

Selon la dernière évaluation des Nations unies, les engagements actuels mènent la planète vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle. Nous savons pourtant qu'au-delà de 2 degrés les conditions mêmes d'existence de l'humanité ne sont pas soutenables.

Cependant, des sources légitimes d'inquiétude demeurent. Nous sommes notamment dubitatifs sur le qui a été donné concernant les objectifs de la France et de l'Union

par la France, elles sont clairement insuffisantes comme l'a pointé le Haut Conseil pour le climat. La récente loi Climat et résilience ou le plan de relance restent trop favorables aux énergies fossiles.

lors que l'on absorbe ailleurs. Cette approche se fonde sur des mécanismes de financiarisation de la nature et laisse cours à toutes les dérives liées aux obligations vertes. On ne peut pourtant pas se satisfaire de simples « droits de polluer Non, planter des arbres à l'autre bout du monde ne diminue pas l'impact des activités des plus gros pollueurs ! Par ailleurs, l'efficacité de ces projets reste à démontrer.

et des États à préserver les biens communs mondiaux, à investir et à faire respecter ces engagements. L'eau, la terre, les forêts et l'air sont des ressources trop précieuses pour les laisser entre les mains de la finance et des multinationales.

importante soit-elle, comment ne pas souligner son aspect dérisoire dès lors que l'industrie pétrolière finance la recherche sur les énergies fossiles à hauteur de 500 milliards de dollars par an ?

lutte pour le climat est aussi une lutte pour l'égalité des droits et donc pour le progrès social partagé. Nous aurions souhaité que le texte mentionne plus clairement la nécessité d'une véritable reconnaissance des droits des peuples autochtones et la priorité donnée à l'humain

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes en état d'urgence climatique. Alors que la COP26 vient de commencer, il est essentiel pour les citoyens du monde entier que nous tenions les promesses de l'accord de Paris. La lutte contre le réchauffement climatique est notre plus grand défi actuel et c'est le plus urgent. Depuis le premier Sommet de la Terre à Stockholm, en passant par les différentes COP qui se sont succédé jusqu'à cette COP26, inquiétudes et déclarations de bonne volonté se sont multipliées. la température de notre planète et les catastrophes environnementales n'ont jamais cessé de s'aggraver. Nous avons connu cette année encore des records de chaleur, des incendies de grande ampleur, des inondations, des canicules et des sécheresses. Le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Le seuil d'une augmentation de température de 1,5 degré pourrait être franchi dès 2030. Le niveau des mers devrait augmenter de près de deux mètres d'ici à la fin du siècle. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je ne fais que reprendre les nouvelles projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publiées le 9 août dernier. La COP26 doit permettre aux pays participants de négocier la mise en oeuvre effective de l'accord de Paris. Les principaux pollueurs ne doivent plus ignorer leurs obligations. L'heure tourne ... Il ne faudrait pas que la COP de Glasgow soit synonyme de douche écossaise ! Les pays doivent s'engager à atteindre des objectifs plus ambitieux pour réduire leurs émissions d'ici à 2030. Ils doivent élaborer des mesures d'adaptation aux conséquences du changement climatique, et naturellement accroître le financement en faveur de la transition écologique. Cela vaut en particulier pour les pays en développement. constate, la situation traîne et les pays peinent à s'accorder sur des sujets clivants, comme la mise en application du marché du carbone. Le président de la COP26, Alok Sharma, a lui-même déclaré qu'il serait difficile de parvenir à un accord, compte tenu de la difficulté des questions à traiter.

de crises migratoires et de nouveaux problèmes sanitaires, comme le paludisme, qui se poseront dans de nombreux endroits de la planète. Je ne connais pas une ville qui ne soit pas affectée par des problèmes de pollution ou de changement climatique.

La France est engagée pour le climat. Nos territoires le sont aussi ! L'échelon local dispose de ressources extraordinaires et d'acteurs concernés, capables de porter des projets territoriaux en faveur de l'environnement et de la biodiversité. L'accord de Paris reconnaît et valorise le rôle des régions, des villes et des autorités locales dans la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne est aussi, naturellement, un acteur clé dans les négociations climatiques. Au fil des ans, elle a adopté une législation environnementale parmi les plus avancées au monde et elle a atteint ses objectifs antérieurs en matière de réduction des émissions. le changement climatique est une menace mondiale, de sorte que les pays européens ne peuvent pas agir seuls. Les Européens ne représentent que 8 % de la population mondiale. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris et l'engagement du président Biden sont venus renforcer nos capacités d'actions, et nous le saluons. De même,

les objectifs de la COP26 doivent nous permettre de ne pas atteindre ces fameux et dramatiques « points de basculement » mentionnés par les experts, c'est-à-dire des changements irréversibles du système climatique. Nous pouvons encore agir. Le groupe centriste votera en faveur de cette proposition de résolution. Il votera pour une coopération ambitieuse vers un nouveau modèle de développement durable, juste et respectueux de l'environnement.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au-delà de l'ambition que nous souhaitons afficher dans ce texte, les enjeux de la COP26 s'inscrivent dans un contexte de « basculement » que nous sommes en train d'effectuer.

L'article 6 de l'accord de Paris prévoit qu'une partie des réductions d'émissions peut être réalisée « des démarches concertées », incluant « l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international », tout en « garantissant l'intégrité environnementale et la transparence

sinon l'espèce humaine ? Il me semble que le concept de biens communs au bénéfice de tous permettra de répondre à l'urgence écologique face à la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes. En somme, l'espèce humaine est-elle capable de s'adapter à elle-même ? Ne sommes-nous pas dans une fuite en avant ? Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la recherche est subventionnée pour travailler sur des programmes de reproduction sélective et développer des lignées d'animaux qui produisent naturellement moins de gaz. La recherche scientifique est-elle une réponse à nos problèmes ? Au-delà de l'activité humaine, ce sont bien nos modes de production qui sont en question. Certains économistes identifient la période que

tout en poursuivant ses investissements dans les hydrocarbures en Arctique, grâce au marché du « droit à polluer ». Tant que nous agirons sur les conséquences du problème au lieu d'en affronter les causes, nous nous enfoncerons dans le réchauffement climatique.

Malgré la décision de Joe Biden de ramener les États-Unis à la table des discussions, cette COP, la vingt-sixième du nom, sera-t-elle la dernière alors que la Russie, le Brésil ou la Chine ne feront pas le déplacement ? Comment ne pas constater que, si l'accord de Paris de 2015 a fait l'objet d'une communication retentissante, les efforts qui ont suivi sont loin d'être suffisants. En effet, la coopération interétatique n'a pas trouvé d'application concrète dans toutes les parties du monde. Signes d'une écologie de façade, les échecs successifs dans l'application concrète de l'accord marquent également le fait que l'écologie est un sujet pris en otage par certains États.

garantir la réciprocité, afin d'éviter que l'enjeu écologique ne soit pris en otage. L'Europe est confrontée à une flambée spectaculaire des prix de l'énergie. Le Gouvernement a récemment adopté une série de mesures Pourtant, ces annonces plus conjoncturelles, voire électoralistes, que structurelles ne font que retarder l'inévitable. En effet, la tension que l'on peut observer sur les marchés de l'énergie jette une lumière crue

L'accord de Paris demeure notre meilleure boussole au coeur de la tempête. En 2015, sa signature marquait un engagement de niveau international. Six ans après, son héritage apparaît bien maigre. Notre ambition est de prendre de l'avance. Il faut demander aux États réticents de se dévoiler. Qui voile la planète, dévoie la France. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant que nous détruisons les conditions de notre survie. Chaque pays doit être comptable de son action. action. Quelles convictions défendons-nous au Sénat ? Tout d'abord, nous prônons l'engagement en action. Cette action ne saurait être confisquée par les idéologies radicales qui ont un autre agenda que celui de la protection de la nature.

de gaz à effet de serre. Outre la route dont l'électrification constitue un enjeu clé, les priorités, en matière de décarbonation des transports, sont connues. Nous devons réaliser un effort considérable de rattrapage sur les infrastructures ferroviaires, accroître la part modale du ferroviaire électrique et développer une politique de fret décarbonée, favoriser le verdissement des flottes de transport de voyageurs et restaurer les équilibres économiques des opérateurs de transport.

Cette COP permettra-t-elle de transcender les égoïsmes nationaux grâce à une coopération internationale largement renforcée ? Nous l'espérons encore. Entre les plaidoyers des « marchés de la peur les partisans de l'écologisme politique, bridant toute initiative technologique ou encore les garants du seul fait compétitif, la voie est étroite, mais elle L'Union européenne, que la France présidera en 2022, représente sur ce point un laboratoire d'exception. Les travaux du Sénat sont comme toujours, en particulier

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « Soit nous stoppons le réchauffement climatique, soit c'est lui qui nous stoppe.

les prévisions antérieures. Plus que jamais, il y a donc urgence à agir réellement et à ne pas se contenter de grandes déclarations. L'accord de Paris de 2015 fixe un objectif commun l'augmentation de la température moyenne de la planète à un niveau inférieur à 2 degrés et la poursuite des efforts pour limiter l'augmentation de cette température à 1,5 degré. Il prévoit également une méthode pour atteindre cet objectif. Les États parties doivent prendre des engagements, actualisés tous les cinq ans, dans la perspective d'un relèvement continu de l'ambition environnementale. À ce stade, la deuxième vague de contributions n'empêcherait pas d'atteindre une hausse des températures d'environ 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle.

l'Union européenne, elle a fixé un nouvel objectif de réduction des émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990, contre 40 % précédemment. Le rehaussement des engagements est l'un des principaux enjeux de la COP26, mais il en existe d'autres comme la question du financement et de l'accompagnement des pays en voie de développement, notamment des pays africains, responsables d'une part infime du réchauffement climatique. Mais au-delà des engagements qui seront, je l'espère, pris à Glasgow, l'essentiel sera de les tenir. Malheureusement, force est de constater que tel n'est pas toujours le cas, tant s'en faut. À cet égard, je constate avec regret que la France est loin d'être exemplaire. Le Haut Conseil pour le climat estime ainsi dans son dernier rapport que les émissions de la France devraient baisser presque deux fois plus vite pour atteindre les objectifs climatiques qu'elle s'est fixés. La récente condamnation de la France par la justice administrative pour son inaction climatique est un autre rappel à l'ordre. Face à cette situation, les parlements, et tout particulièrement notre assemblée, doivent veiller au respect des engagements pris. Nous ne devons pas laisser les nombreuses associations, les ONG ou la justice jouer le rôle de vigie des engagements gouvernementaux en matière d'environnement.

Vous l'aurez compris : au-delà du caractère crucial de cette COP, le plus important sera ensuite de maintenir le cap pour atteindre les objectifs fixés. C'est un travail que nous devons mener au quotidien en tant que parlementaires, mais aussi en tant que citoyens. La parole

du mur. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, à l'exception de l'année 2020, durant laquelle la covid-19 a entraîné une baisse de 6 % des émissions mondiales. Chaque année, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, les températures grimpent et les événements extrêmes sont de plus en plus fréquents. L'année 2021 est une année importante, puisqu'elle aura été marquée par le congrès mondial de l'UICN, la COP15 pour la biodiversité et la COP26. Je regrette d'ailleurs que ces rassemblements internationaux soient distincts, tant la dégradation de la biodiversité, le réchauffement climatique et la désertification sont

Cette proposition de résolution sénatoriale en est aussi la preuve. Le Parlement est pleinement investi dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment au travers de l'élaboration de politiques d'adaptation : nous devons « conserver ce qui vaut et adapter ce qu'il faut.

Il nous faut une stratégie en la matière ! Les énergies renouvelables doivent être développées, mais nous ne pourrons pas nous passer du nucléaire, qui fait partie de la solution, n'en déplaise à certains. Le nucléaire est reconnu par le GIEC comme une solution indispensable pour respecter les accords de Paris. Limiter le réchauffement climatique n'est pas hors d'atteinte. Cela suppose d'entamer une révolution énergétique globale et de prévoir des transitions dans tous les pans de notre économie. Selon le rapport du GIEC, il existe de nombreuses possibilités de lier cette atténuation et cette adaptation à l'atteinte d'autres objectifs sociétaux, grâce à des approches globales. Pour que les efforts déployés soient fructueux, il faut se doter d'outils appropriés, de structures de gouvernance adaptées et il faut renforcer notre capacité de réaction.

de tenir nos promesses et de ne pas en formuler d'autres si nous ne sommes pas capables de les tenir- cela vaut également pour le débat national. De plus, il faut finaliser les règles de mise en oeuvre du pacte sur le climat, notamment au sujet de la transparence, c'est-à-dire la façon dont les États rendent compte de leurs actions et de leurs résultats.

Saisissons-la, à l'occasion de cette COP26 ! Saisissons aussi l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour donner une nouvelle impulsion. Malheureusement, cette présidence sera partiellement paralysée par l'élection présidentielle.

leur engagement budgétaire, pour atteindre 11 milliards d'euros d'ici à 2024. C'est évidemment un signal très positif. De plus, la COP26 offrira l'occasion de confirmer la prise de conscience croissante du lien entre climat et biodiversité.

instants. La séance est suspendue. La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici aujourd'hui à l'aboutissement d'un travail collectif et, si vous me permettez l'expression, d'une belle aventure parlementaire. Voilà près de deux ans, déjà, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable lançait une mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique. Six mois plus tard, en juin 2020, la mission publiait un rapport inédit, constatant le risque d'un accroissement de la pollution numérique. Si rien n'est fait, le secteur pourrait représenter 7 % de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2040. Notre objectif était clair : agir sans attendre, pour combler un angle mort de nos politiques environnementales et prendre le tournant de la transition numérique, tout en s'assurant que ce secteur, au demeurant indispensable à la transition écologique, ne devienne pas la source d'une pollution exponentielle. En octobre 2020, nous déposions avec de nombreux collègues, dont Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte et Hervé Maurey, une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, dite REEN, retranscrivant les propositions de notre rapport. En commission, en décembre, puis en séance publique, en janvier, nous avons amélioré et complété ce texte, qui est ainsi passé de 24 à 31 articles. Je voudrais remercier les collègues de l'ensemble des groupes politiques qui ont participé à cet enrichissement : ce texte, soutenu à l'origine par certains d'entre nous, est sans aucun doute devenu celui de l'hémicycle tout entier, au terme d'un travail collectif dont nous pouvons nous féliciter. Je tiens tout particulièrement à remercier Hervé Maurey, qui présidait la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au moment du lancement de nos travaux, et mes deux collègues rapporteurs, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, avec lesquels j'ai travaillé étroitement pour améliorer le texte. Mes remerciements vont également au président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Jean-François Longeot, qui n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la poursuite de la navette. Je salue également Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, qui a contribué à enrichir la proposition de loi. Je veux aussi remercier les collaborateurs et administrateurs qui m'ont accompagné dans un climat de confiance permanent. Mais, une fois n'est pas coutume, je tiens aussi à vous remercier particulièrement, monsieur le secrétaire ? ... ainsi que votre cabinet, pour les échanges constructifs dans un climat de sincérité que nous avons pu entretenir tout au long de ce parcours. Le texte transmis à l'Assemblée nationale comptait 31 articles. Il a été adopté par les députés à l'unanimité le 10 juin C'est ce texte modifié, comptant désormais 36 articles, que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a examiné le 20 octobre. L'Assemblée nationale a globalement conforté le travail que nous avons effectué en première lecture. Je salue à cet égard le rapporteur, Vincent Thiébaut, et le rapporteur pour avis, Éric Bothorel, pour leur sens de l'écoute et leur sérieux, mais aussi pour leur appropriation du sujet et de ce texte. Nous regrettons néanmoins certains choix arrêtés en première lecture par l'Assemblée nationale et par le Gouvernement. Je commencerai par la suppression de l'article 23 relatif à la collecte de données environnementales par l'Autorité

Malheureusement, le Conseil constitutionnel, en censurant cet article dans sa décision sur ladite loi, nous a donné raison. Ce sujet nous semblait toutefois trop important pour être abandonné. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi à article unique reprenant l'article censuré par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de la deuxième qui nous est soumise aujourd'hui. Examinée en première lecture, conjointement à l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi REEN, elle est totalement complémentaire de ce dernier texte, dont elle facilitera l'application, en armant pleinement le régulateur dans la mise en place d'une régulation environnementale du secteur numérique.

Au-delà de ce sujet, nous regrettons le recul global de l'ambition de la proposition de loi REEN à l'Assemblée nationale : nous sommes convaincus que nous aurions pu être plus audacieux et innovants. Le texte, tel que l'ont modifié les députés et le Gouvernement, est imparfait et incomplet, et cette deuxième lecture a, je ne vous le cache pas, un petit goût d'inachevé. Je ne ferai pas la liste des points de désaccord persistants ; je laisserai les rapporteurs les présenter plus en détail. Il m'est impossible, toutefois, de ne pas aborder la question de la rémunération pour copie privée, à l'article 14 B.

dont plusieurs dispositifs visaient justement à renforcer la compétitivité du réemploi aux dépens du neuf. Très bien ! La confusion entretenue par le Gouvernement entre les difficultés conjoncturelles rencontrées par le monde de la culture dans le contexte de la crise sanitaire et la dimension structurelle du financement par la rémunération pour copie privée est particulièrement dommageable. Nous espérons, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous annoncerez aujourd'hui des mesures de compensation pour le secteur des équipements Ce constat étant fait, la question qui s'est posée aux deux rapporteurs du texte et à moi-même, était de savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis de cette proposition de loi REEN.

Trois raisons nous semblent justifier cette stratégie. Premièrement, certains reculs de l'Assemblée nationale, notamment sur la rémunération pour copie privée, ne doivent pas occulter les avancées profondes et nombreuses permises par la proposition de loi, qui ne constitue que la première pierre à l'édifice de la régulation environnementale du numérique dans notre pays. Si nous l'adoptons, ce texte placera la France dans une position de précurseur sur la scène européenne en matière de transition environnementale du numérique, ce qui lui permettra de défendre ce sujet avec force et crédibilité dans les négociations avec les États membres de l'Union européenne. Deuxièmement, si nous l'adoptons, la proposition de loi REEN produira des effets très rapidement, d'autant

Soyons clairs : si nous amendons aujourd'hui le texte qui nous est soumis, il est peu probable qu'il soit transmis en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Les points de désaccord avec le Gouvernement sont réels ; ils sont parfois importants, comme sur la rémunération pour copie privée. Je pense toutefois qu'ils sont minoritaires et qu'ils ne justifient pas de sacrifier la majorité des dispositions que nous pourrions voir entrer dans le droit avec un vote conforme. Voilà, mes chers collègues, la voie que je vous propose de suivre aujourd'hui. Elle n'est pas pleinement satisfaisante, j'en conviens. Mais sachons également nous réjouir de ce que nous avons fait en ce moment où la planète planche à Glasgow pour la COP26, le Sénat a fait oeuvre utile en plaçant la France en position de pionnière en matière de transition numérique durable. Je note d'ailleurs que notre proposition de loi a déjà produit ses effets. Depuis son dépôt en octobre 2020, la question de l'empreinte environnementale du numérique s'est totalement imposée dans le débat public, au point que de nombreux acteurs, notamment les opérateurs mobiles, ont commencé à engager des actions concrètes. Je forme donc le voeu que vous suiviez la commission dans sa stratégie, pragmatique et responsable, d'adoption conforme de la proposition de loi REEN.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, aux côtés de mon collègue corapporteur Guillaume Chevrollier, pour examiner la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, en deuxième lecture, et la proposition de loi visant à renforcer la régulation de l'environnement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), en première lecture. Je vais vous présenter ces deux textes, que notre commission a adoptés sans modification. Commençons par la proposition de loi REEN. Je rappelle que le texte que nous avions transmis à l'Assemblée nationale en janvier dernier comptait 31 articles répartis selon cinq axes faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact environnemental ; limiter le renouvellement des terminaux, principaux responsables de l'empreinte carbone du numérique ; promouvoir le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux aller vers des centres de données et des réseaux moins énergivores ; promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Les députés ont en grande partie conforté le travail du Sénat. Nombre de nos apports ont en effet été conservés, notamment : la création d'une formation de sensibilisation à l'impact environnemental du numérique et à la sobriété numérique dans l'enseignement primaire et secondaire, qui fait l'objet de l'article 1 le renforcement du délit d'obsolescence programmée prévu à l'article 6 et son extension à l'obsolescence logicielle prévue à l'article 7. L'Assemblée nationale a même introduit de nouvelles dispositions, conformes à l'objectif et à l'esprit de la proposition de loi initiale. J'en citerai trois : la mise en place d'opérations de collecte nationale d'équipements numériques, accompagnées d'une prime au retour, à l'article 12 A ; la suppression de l'obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables, à l'article 14 ; le le renforcement des prérogatives du maire en matière de déploiement d'infrastructures de télécommunications, à l'article 23 A, et de suivi des investissements réalisés par les opérateurs en faveur du partage d'infrastructures, à l'article 23 B. Bien sûr, nous déplorons également certains reculs opérés à l'Assemblée nationale sur des sujets structurants, par exemple : la suppression de l'allongement à cinq ans de la durée de la garantie légale de conformité, à l'article 11, et de la durée de réception des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien, à l'article 9 ; la suppression du caractère contraignant du référentiel d'écoconception des services numériques, que nous souhaitions imposer aux fournisseurs de tels services, à l'article 16. Ces quelques réserves ne doivent pas occulter les avancées profondes permises par ce texte, que nous vous proposons d'adopter conforme. Faisons oeuvre utile en permettant aux nombreuses dispositions de la proposition de loi d'entrer en vigueur Je terminerai en évoquant succinctement la proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Arcep, qui vise à armer pleinement le régulateur dans la mise en place d'une régulation environnementale du secteur numérique et à faciliter l'application de la proposition de loi REEN. Ce texte parfaitement consensuel pourrait être examiné à l'Assemblée nationale au mois de décembre prochain, ce qui lui permettrait d'entrer en vigueur dans les meilleurs délais. Enfin, pour conclure, et conformément à ce que disait précédemment Patrick Chaize, cette proposition de loi, en révélant une problématique jusqu'à présent ignorée, celle de l'impact environnemental du numérique, a fait l'effet d'un électrochoc. Une large sensibilisation s'est en effet opérée et, déjà, un bon nombre d'acteurs se sont engagés dans des actions de réduction de leur empreinte ou des campagnes de collecte de terminaux. Il est donc urgent de traduire dans la loi l'ensemble des dispositions qui figurent dans la proposition de loi qui vous est soumise. La parole

le principal auteur de la proposition de loi, Patrick Chaize : l'article 14 B, relatif à la rémunération pour copie privée sur les équipements reconditionnés, et l'article 15, relatif à la lutte contre le démarchage téléphonique. Commençons par la rémunération pour copie privée. Pour rappel, celle-ci est une contribution prélevée sur les supports d'enregistrement- CD et DVD vierges, mémoires et disques durs d'ordinateur, de téléphone ou de tablette -permettant de compenser la perte subie par les artistes en raison du développement de la possibilité de copier leurs oeuvres. Au moment de la rédaction de la proposition de loi, la rémunération ne s'appliquait qu'aux produits neufs lors de leur mise en circulation. Au stade de l'examen du texte en séance publique, en première lecture, nous avions appris que la commission pour la rémunération de la copie privée avait engagé une réflexion tendant à assujettir également les appareils reconditionnés. Après nous être assurés qu'une exonération des biens reconditionnés ne retirerait pas de ressources au monde de la culture, mais ne ferait que la priver d'une recette supplémentaire et hypothétique, nous avions adopté un amendement créant un article 14 B visant à exonérer du paiement de la rémunération les appareils y ayant été assujettis une première fois, afin de renforcer la compétitivité des équipements Malheureusement, le 1 juin dernier, la commission pour la rémunération de la copie privée a permis l'application d'un barème de la rémunération pour copie privée sur les biens reconditionnés à compter du 1 juillet 2021. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter en séance publique un amendement de réécriture de l'article 14 B, venant entériner la décision de la commission précitée. Nous regrettons vivement ce choix qui tend à revenir sur l'exonération votée au Sénat. D'autres choix étaient possibles, plusieurs pays ayant choisi d'exonérer intégralement les biens reconditionnés ou de ne taxer que les équipements qui n'ont pas déjà fait l'objet de prélèvements quand ils quand ils étaient neufs. Si nous ne pouvons donc qu'être vivement défavorables au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, nous nous réjouissons toutefois de l'application d'un taux spécifique et réduit pour les équipements reconditionnés, ainsi que de l'exonération des acteurs de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais maintenant évoquer un deuxième point d'attention à l'article 15 , introduit par l'Assemblée nationale. Dans l'ensemble, nous accueillons favorablement cet article qui vise à lutter contre le démarchage téléphonique abusif au travers de l'encadrement des automates d'appels et des conditions de territorialité des identifiants issus du plan de numérotation national. Avant l'examen du texte en commission, certains acteurs nous ont toutefois fait part d'inquiétudes s'agissant d'effets indésirables que le dispositif pourrait induire pour les entreprises ayant recours à des automates d'appels pour la gestion des relations client. Après avoir mené l'enquête, ces inquiétudes ne nous semblent pas fondées. En effet, l'article 15 vise spécifiquement à lutter contre l'usurpation d'identifiant, particulièrement usitée pour les canulars et arnaques téléphoniques. d'une part, il s'inscrit dans la continuité du droit actuel qui interdit déjà le recours aux numéros mobiles et aux numéros masqués pour les centrales d'appels il n'aura pas pour conséquence de proscrire l'utilisation d'identifiants géographiques ou non géographiques par les centres d'appels, mais uniquement de leur réserver certaines tranches de numéros, afin de faciliter l'authentification de l'appelant. Ces éléments ont permis de rassurer les acteurs concernés. En tout état de cause, nous serons particulièrement attentifs à ce qu'il n'y ait aucun effet de bord. Si tel était le cas, le Gouvernement s'est engagé à ce que de tels effets soient corrigés par voie réglementaire.

Si les débats ont été vifs, c'est que le sujet est d'importance, et je me félicite que la représentation nationale- ici, au Sénat, comme au Palais Bourbon -s'en soit pleinement saisie. Je tiens à saluer le travail des rapporteurs, et tout et tout particulièrement celui, approfondi, utile et riche du sénateur Patrick Chaize, qui est à l'origine de ce texte et grâce auquel nous sommes aujourd'hui à même de mettre en oeuvre des mesures qui auront un impact tangible sur la vie de nos concitoyens.

général. Je ne suis pas toujours d'accord avec le sénateur Patrick Chaize, et c'est heureux, mais je voudrais encore une fois, et très personnellement, le remercier de la qualité du dialogue que nous avons eu et de la richesse du travail effectué.

Une fois n'est pas coutume, je souhaite commencer mon propos non par un sujet transcendant, mais en mettant l'accent sur les mesures concrètes que vous allez examiner et, je le souhaite, adopter aujourd'hui. Je ne détaillerai pas toutes les mesures de ce texte, mais seulement quelques-unes,

L'article 6 de la proposition de loi prévoit ainsi de simplifier la définition de la lutte contre l'obsolescence programmée, en particulier logicielle, pour faciliter la lutte contre celle-ci et ainsi rendre possibles les poursuites, voire les condamnations, qu'appellent de leurs voeux les associations de défense des consommateurs. Les articles 1, 1 et 2 font le pari de la formation et de la sensibilisation des jeunes et des étudiants pour que ce qui apparaît aujourd'hui comme exotique- l'écoconception, notamment -devienne demain la norme, en pratique et dans les esprits. Les articles 14 AA et 14 permettent, par des mesures concrètes- la mise à disposition d'informations et l'obligation de fournir des pièces détachées aux reconditionneurs -d'allonger la durée d'utilisation des terminaux, ce qui est un gain en termes, à la fois, de pouvoir d'achat et d'environnement. L'article 23 A, en encadrant le partage des pylônes en zone rurale, contribue à la rationalisation des infrastructures de réseaux sur le territoire français et améliore ainsi la connectivité pour nos concitoyens, avec un impact environnemental optimisé. Je tiens à signaler, par ailleurs, qu'il s'agit de répondre à une demande des collectivités territoriales pour lutter contre la spéculation foncière liée au déploiement des pylônes en zone rurale. Je pourrais citer bien d'autres mesures de cette proposition de loi qui, comme celles-ci, sont à la fois très concrètes et avec un fort impact. Car c'est la caractéristique de ce texte et, plus globalement, de la politique du Gouvernement que de faire le choix du pragmatisme, des petits pas, parfois, mais toujours dans la bonne direction, plutôt que des déclarations à l'emporte-pièce. Ce pragmatisme est au coeur de la stratégie nationale pour le numérique et l'environnement que je défends avec la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l'économie, des finances et de la La feuille de route interministérielle que nous avons construite ensemble, et rendue publique en février 2021, a ainsi pour objectif de faire converger les transitions écologique et numérique au travers de trois axes que je tiens à rappeler ici. Le premier axe, c'est la connaissance de l'empreinte environnementale du numérique. Il est en effet aujourd'hui nécessaire d'apporter des données précises et objectives sur les impacts positifs et négatifs de l'ensemble du cycle de vie des services numériques sur l'environnement. Cette approche doit être multicritère et intégrer aussi bien la dimension des émissions de gaz à effet de serre que la consommation d'énergie, d'eau et de ressources en matières premières. Le second Le second axe, c'est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en tant que telle. Alors que les projections montrent une croissance importante des usages numériques, il s'agit de maîtriser, voire de réduire, l'empreinte environnementale du numérique, liée à la fabrication des équipements et terminaux et aux usages. Le troisième et dernier axe, c'est la mobilisation du numérique au service de la transition écologique. Le numérique permet déjà d'optimiser la consommation d'énergie, de réduire nos trajets, d'éviter ou de mieux gérer des déchets. Il s'agit désormais de s'appuyer sur le potentiel du numérique pour accélérer la transition écologique. proposition de loi, qui fait l'objet d'une discussion commune, reprend dans un article unique les dispositions agréées par les deux chambres à l'issue de la navette parlementaire, visant à la création d'un pouvoir de collecte de données environnementales

dans la première proposition de loi du sénateur Chaize. Il s'agit d'un outil stratégique permettant, de manière inédite, à l'Arcep de collecter des données sur l'ensemble des acteurs du numérique et non plus seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, auprès des seuls opérateurs télécoms. En réintroduisant cette disposition qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel au regard de sa doctrine en matière de cavalier législatif, vous ferez un acte utile. Il s'agit bien, en effet, de pallier des difficultés juridiques et techniques, et ainsi de restaurer la pleine portée opérationnelle de la première

Tout se passe comme si, comme le dit Ferghane Azihari dans une interview récente au magazine, « le progrès était systématiquement vu par certains d'entre nous comme source de corruption et de décadence Je le dis très honnêtement, si nous continuons ainsi, nous allons dans le mur. Le combat environnemental se meurt d'un antilibéralisme qui ne lui est consubstantiel qu'en France. une fois, cela nous envoie dans le mur pour une raison assez simple. Sur cette planète, un humain sur trois vit avec moins de 3 dollars par jour. La population mondiale continuera à augmenter, quoi que nous fassions. Les ressources, énergie et matières premières, sont limitées. Une partie de cette tension, qui est d'ordre mathématique, peut être résolue par une modification de la consommation.

Merci Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis que le Sénat replace le numérique et l'écologie au centre de ses préoccupations, en proposant un texte ambitieux et équilibré. En revanche, je regrette que, une fois passé devant l'Assemblée nationale, le texte ait perdu quelque peu de sa substance. Il n'en demeure pas moins que la France est le premier pays européen à légiférer sur ce sujet. Nous encourageons les autres États membres à nous suivre. La transformation numérique de notre société nous oblige à une certaine exigence, compte tenu des enjeux écologiques actuels. La technologie et le progrès technique nécessitent de transformer nos modèles de production, de croissance et de consommation en raison de leur impact négatif sur l'environnement. D'après les travaux de la mission d'information, si rien n'était fait, le secteur du numérique serait en 2040 de l'émission de 24 millions de tonnes d'équivalent carbone, soit environ 7 % des émissions de la France. Le secteur des nouvelles technologies représente à lui seul entre 6 % et 10 % de la consommation mondiale d'électricité. Le numérique nous invite donc à explorer les chemins de la transition écologique en prenant en compte les dimensions sociales et collectives de cette évolution. Certaines associations fournissent un travail important pour introduire la problématique de l'empreinte environnementale du numérique dans le débat public. Nous sommes tous et toutes concernés. Acteurs privés comme publics, nous devons nous responsabiliser sur ce sujet. C'est pourquoi l'article 1 du texte incite à la sobriété numérique. En effet, un travail de pédagogie doit être mis en place pour enfin apprendre à se déconnecter.

aux équipements mobiles usés et remis en état. Cette disposition dénature le texte sur ce point précis. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si je salue l'objectif initial de cette proposition de loi, je ne peux qu'encourager à davantage d'efforts dans l'élaboration d'une véritable politique environnementale du numérique. La

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique que nous examinons aujourd'hui a été adoptée à la quasi-unanimité dans cet hémicycle en janvier 2021, puis à l'Assemblée nationale en juin dernier. Ce texte de consensus - je salue d'ailleurs particulièrement le travail de mes collègues Jean-Michel Houllegatte, Guillaume Chevrollier et Patrick Chaize Chaize -, fruit d'un travail de fond mené par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, répond en effet à l'urgence d'interroger, de mesurer et d'évaluer l'empreinte environnementale du numérique pour mieux la réduire, dans la perspective d'un développement soutenable, pour faire du numérique un accélérateur vertueux de la transition écologique. L'évolution significative des usages, des moyens, des outils, et la montée en puissance de la 5G rendent le sujet incontournable. Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'esprit du texte et ses objectifs ont été préservés, et les mesures emblématiques que nous avions adoptées ont été respectées. Nous déplorons néanmoins la suppression de certaines initiatives sénatoriales. Ces modifications dénotent peut-être une relative frilosité des députés, qui aboutissent finalement à un texte cohérent, mais un peu moins ambitieux. Parmi les suppressions regrettables - j'en mentionnerai quelques-unes -, il y a évidemment celle de l'intégration de l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE (responsabilité Personnellement, j'ai toujours envie de mettre en avant la responsabilité sociétale des organisations (RSO), qui me paraît particulièrement intéressante concernant ce sujet.

Qu'il s'agisse du secteur public ou privé, tous les acteurs sont appelés à participer à une évolution favorable sur cette problématique. Nous regrettons également la suppression du crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, qui visait essentiellement à encourager l'évolution de leur approche du numérique vers plus d'efficience et, encore une fois, vers plus de sobriété. La suppression de l'intégration de l'impact environnemental du numérique dans le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables Cette mesure défendue par un amendement de notre groupe ambitionnait de faire de l'achat public un levier significatif pour réduire l'empreinte carbone du numérique, en inscrivant ainsi la politique d'achat dans une démarche de durabilité des produits et un usage plus raisonné des ressources.

Saluons notamment l'ajout de quelques dispositions, de portées parfois inégales, qui rejoignent les objectifs généraux que nous nous étions donnés. Je soulignerai notamment la formation à l'impact environnemental du numérique dans l'enseignement supérieur, qui offre des perspectives d'avenir pour éduquer les jeunes générations, et modifier à terme les pratiques en faveur d'un plus grand respect de notre environnement. À l'échelle de nos territoires, notons également l'ajout de la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les dossiers d'information Enfin, ce texte conserve également - et nous nous en réjouissons -, au chapitre V, créé sur l'initiative de notre groupe, l'objectif de promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires à travers en particulier deux articles. Le premier vise à mieux intégrer les dans les systèmes énergétiques locaux dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux. prévoit que les collectivités de plus de 50 000 habitants compléteront leur rapport sur leur situation en matière de développement durable par la présentation d'une stratégie numérique responsable. Cette proposition de loi, malgré les limites que je viens d'évoquer, affiche donc une première ambition essentielle : faire du numérique un accélérateur de la transition écologique à l'empreinte environnementale soutenable. Elle conforte les démarches d'évaluation environnementale dont les politiques de développement durable ne peuvent se départir et une réflexion appuyée sur des indicateurs, des données objectives, qui permettent une meilleure régulation de l'ensemble de la chaîne numérique. Notre proposition vise à créer les conditions d'une progression collective fondée sur une meilleure information et sur la responsabilisation des acteurs et des usagers.

C'est une responsabilité sociétale que nous défendons. Elle est bien sûr construite avec les usagers, mais également avec nos territoires, qui constituent l'indispensable maillon garantissant l'équilibre entre transition numérique et transition écologique, permettant d'harmoniser les attentes légitimes liées au déploiement d'une couverture numérique ambitieuse et le respect des enjeux climatiques. Le Sénat s'est montré pionnier sur ce sujet, il faut le souligner. Faisant notamment écho aux rapports et aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, de l'Arcep, du Haut Conseil pour le climat concernant l'empreinte environnementale de la 5G, il a démontré, une nouvelle fois, sa capacité à faire émerger dans le débat national des problématiques essentielles pour les citoyens et les territoires, à accélérer les prises de conscience et à les traduire en solutions Cette proposition de loi constitue une première étape pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Elle répond au besoin d'engager un débat ambitieux, et ouvre une voie sur laquelle nous continuerons de travailler. C'est dans ce sens que nous voterons ce texte. Le numérique ne doit pas dégrader la situation actuelle, il doit nous conduire à la société décarbonée de demain. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, contrairement aux idées reçues, le numérique n'est pas immatériel. Il a bien un visage, une odeur, un son, un poids et surtout un coût pour notre environnement. Le traitement d'une requête sur un moteur de recherche mobilise des ressources matérielles, un smartphone, une box internet, des routeurs, un pare-feu, des équipements réseau, un serveur, des câbles sous-marins et des centres de données. Les centres de stockage de données, qui sont en effet responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique, cherchent des solutions. Le de type adiabatique peut être une de ces solutions. Le centre que j'ai visité en mars dernier à Saint-Ouen-l'Aumône n'utilise pas de climatisation et consomme entre 40 % et 50 % d'énergie en moins La chaleur dégagée par les machines est mélangée à l'air extérieur et réutilisée pour refroidir les ordinateurs. Des solutions existent bien, mais elles sont encore expérimentales et ne sont pas encore à la hauteur du coût du numérique qui engendre entre 4 % et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, chiffres qui ne sont pas près de décroître. Alors que débute le sommet de la COP26, le Gouvernement et les parlementaires de tout bord se mobilisent pour faire du numérique un levier de la transition écologique. Cette proposition de loi qui arrive en seconde lecture au Sénat en est le témoignage, et elle comporte de réelles avancées. Des mesures concrètes pourront voir le jour très prochainement. Je pense notamment à la prise de conscience, par les usagers, de l'impact environnemental du numérique, la souscription d'engagements contraignants des opérateurs de réseau auprès de l'Arcep, à la suppression de l'obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables, au droit à la réversibilité des mises à jour, ou encore à la promotion de centres de données et de réseaux moins énergivores. Alors certes, et cela a été dit, le texte que nous nous apprêtons à voter est en deçà des attentes. Un certain nombre de dispositifs ont été supprimés par l'Assemblée nationale. Il s'agit du prix à payer pour la coconstruction entre parlementaires, acteurs privés et Gouvernement. ce texte, il s'agit non pas de se faire plaisir pour exister, mais bien d'avancer ensemble en faveur de la transition écologique du numérique. Des mesures radicales, mal acceptées par les opérateurs, n'auraient sans doute eu aucun effet. De ce fait, j'en profite pour saluer l'expertise, l'esprit pragmatique et positif de l'auteur de cette proposition de loi, Patrick Chaize, et de ses rapporteurs. Enfin, notre travail doit s'articuler avec les mesures complémentaires du Gouvernement. Je fais référence à la feuille de route qui permettra d'actionner quinze mesures fortes, comme l'ambition pour l'État d'acheter 20 % de matériel informatique, de téléphones fixes et portables reconditionnés. transition écologique) mènent une mission conjointe pour identifier et évaluer les facteurs permettant de quantifier l'empreinte environnementale des réseaux. L'étude est en cours, et les résultats seront publiés en 2022. Cette mission s'articule d'ailleurs parfaitement avec la proposition de loi annexe qui vise à donner à l'Arcep le pouvoir de recueillir des données sur les impacts environnementaux des services de communications électroniques. Notre prise de conscience est certes tardive, mais elle est bien réelle. Face à la croissance exponentielle de nos usages numériques, nous ne pouvions plus regarder passer les trains sans agir. Ce texte doit donc être considéré comme un premier pas décisif pour que nous puissions enfin faire émerger un numérique durable et responsable face aux enjeux climatiques.

Le numérique doit être envisagé comme un avantage dans la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. Il sera d'une importance capitale dans de nombreux secteurs de nos vies, par exemple dans l'agriculture ou encore

je me réjouis que nous ayons à examiner en seconde lecture la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat le 12 janvier dernier. Il est en effet assez rare que les propositions émanant du Sénat soient reprises et votées, à l'unanimité également, à l'Assemblée nationale.

Face aux occasions offertes par le secteur du numérique et devant le formidable horizon que ces nouvelles technologies ouvrent, la question de l'empreinte environnementale est bien souvent occultée. Avec cette proposition de loi, la France devient un des pays précurseurs dans ce

En première lecture, le travail des deux rapporteurs, nos collègues Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, avait permis d'enrichir fortement le texte. Je me réjouis de voir qu'une grande partie des mesures adoptées au Sénat ont été conservées à l'Assemblée nationale. L'instauration d'un observatoire des impacts environnementaux du numérique paraît en effet indispensable pour permettre à la France de poursuivre la réflexion sur ce sujet. Le renforcement du délit d'obsolescence programmée et son extension à l'obsolescence logicielle, de même que le droit à la désinstallation des mises à jour non nécessaires me paraissent également pertinents et nécessaires. À l'heure où la durée de vie moyenne d'un smartphone est de vingt-quatre mois, cette législation permettra aux utilisateurs de renouveler leur smartphone ou leur tablette par besoin et non par obligation.

d'une plus grande réutilisation des équipements numériques et de les assujettir à une redevance qui ne devrait concerner que les équipements neufs. C'est contraire à l'esprit de la proposition de loi. Certes, un taux spécifique et réduit s'appliquera pour les équipements reconditionnés,

À la veille du déploiement de la 5G et de la multiplication des antennes relais, ces mesures vont dans le bon sens, mais ne me paraissent pas suffisantes. Il est important de redonner aux maires la maîtrise de l'aménagement du territoire dont ils ont la responsabilité. Compte tenu du calendrier législatif, nous avons fait le choix de voter ce texte conforme

de le voir progresser vers une adoption, sachant qu'il n'existe à ce jour aucune législation robuste permettant de contrôler, de réguler ou de réduire les dommages indéniables du numérique, tel qu'il se pratique aujourd'hui, Ignorée, minimisée, absente du débat public voilà encore peu, l'empreinte environnementale du numérique est devenue un sujet incontournable La durabilité et la sobriété, qui doivent être au coeur de la notion d'écoconception, ne peuvent plus être esquivées par les acteurs du numérique. À la veille de la présidence française de l'Union européenne, ce texte est un premier jalon. Alors que le numérique est affiché comme l'une des priorités majeures de cette présidence, cette proposition de loi peut être une étape significative. En première lecture, nous avons salué le renforcement des orientations de la proposition de loi sur plusieurs volets : lutte contre l'obsolescence programmée, qui n'a pas obtenu, jusqu'ici, les résultats escomptés ; soutien aux activités de reconditionnement, capital pour contrer la spirale du renouvellement permanent de nos terminaux ; obligation de l'écoconception ; empreinte environnementale des réseaux et centres de données ; et promotion de stratégies numériques responsables sur les territoires, car rien n'est solide ni efficace s'il ne se décline concrètement sur nos territoires. Le chemin parcouru est donc satisfaisant. Demeurent cependant plusieurs frustrations et soucis dont plusieurs d'entre vous se sont déjà fait l'écho. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale n'a pas toujours correspondu à la hauteur des enjeux soulevés au départ. Des dispositions structurantes ont vu leur portée réduite, quand elles n'ont pas été supprimées : l'assujettissement des biens reconditionnés à la rémunération pour copie privée et le référentiel de l'écoconception des services numériques sont nos deux principaux problèmes, sans oublier la suppression de l'allongement de la garantie légale de conformité de la durée des mises à jour.

Le coût supplémentaire risque d'être dissuasif pour les consommateurs, qui se dirigeront vers du neuf bas de gamme ou du reconditionné importé au bilan carbone déplorable. Est-ce vraiment l'esprit du texte que nous voulions voter ?

jusqu'en juillet 2022 et limiter le taux à 1 %. Tel est l'objet de deux de nos amendements. Mme la ministre Roselyne Bachelot avait promis des dispositifs de soutien consistants pour le secteur du reconditionnement ; nous les attendons toujours. Il est donc important d'avoir ce débat aujourd'hui et d'interpeller le Gouvernement,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai bien conscience que l'option majoritairement retenue ici est d'aboutir à un vote conforme,

Et pourtant, il nous est apparu que ce texte aurait pu être très sensiblement amélioré sans nécessairement en modifier l'économie globale.

que l'affichage de grandes ambitions publiques de régulation a parfois constitué un atout pour le développement de notre économie. Il ne s'agissait pas du numérique à l'époque, mais de l'électronique. C'est pourquoi je m'étonne que l'obligation de l'écoconception des sites ait été transformée en une simple invitation à bien faire. Certes, ce n'est pas non plus une invitation à mal faire, mais cette disposition paraît très raisonnablement peu ambitieuse. Ce dispositif de régulation, réécrit de manière à instituer de vrais référentiels opérationnels, c'est-à-dire standardisés, évolutifs et par catégorie de services numériques, aurait permis de contribuer grandement à la protection de l'environnement.

demain. La régulation environnementale est un moyen de favoriser l'accessibilité sociale des outils numériques. Il faut donner à chacune et à chacun, c'est-à-dire à tout le monde, les moyens d'être écologiste.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, en deuxième lecture, est l'aboutissement des travaux de la mission d'information mise en place en 2019, sous la houlette de Patrick Chaize et Jean-Michel Houllegatte, par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Ses travaux ont notamment permis de se pencher, pour la première fois, sur l'impact environnemental du numérique en France et d'élaborer un certain nombre de préconisations, reprises dans cette proposition de loi dont j'ai l'honneur d'être coauteur. Nous pouvons nous féliciter que texte ait été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, dans une version qui maintient en grande partie les apports de notre assemblée. Cela confirme, s'il en était besoin, que le Sénat n'est pas toujours à la traîne de l'Assemblée nationale en matière environnementale et qu'il n'est pas l'assemblée caricaturale que l'on veut parfois présenter Les députés ont ainsi conservé, voire conforté, un certain nombre de dispositions relatives à la sensibilisation des utilisateurs, à la limitation du renouvellement des terminaux, à l'efficience énergétique des centres de données et des réseaux et à la mise en oeuvre de stratégies numériques responsables au niveau local. Si nous pouvons nous réjouir que l'Assemblée nationale ait validé de nombreuses positions du Sénat, certaines modifications apportées par les députés sont regrettables, car en retrait par rapport à l'ambition exprimée par notre assemblée.

L'allongement à cinq ans de la durée de la garantie légale de conformité ainsi que les différentes dispositions visant à créer la confiance et à rendre plus attractifs les produits reconditionnés ont été supprimés. l'application de la rémunération pour copie privée aux produits reconditionnés, adoptée par l'Assemblée nationale, va avoir tendance à réduire la compétitivité de ces derniers- c'est une évidence. Ces mesures sont perçues par de nombreux acteurs comme un nouveau recul du Gouvernement dans le domaine de l'économie circulaire. À cet égard, je rappellerai que les crédits du fonds de réparation et de réemploi, créé par le Sénat dans le cadre de la loi AGEC, ont été revus à la baisse de manière draconienne, au point de remettre en cause l'existence même de ce fonds. Certaines mesures relatives à la promotion d'usages durables numériques ont également vu leur portée diminuée, l'Assemblée nationale ayant, dans certains cas, préféré l'incitation à l'obligation. C'est le cas notamment de l'information sur les émissions de la vidéo à la demande, que le Sénat avait adoptée sur ma proposition. Compte tenu des contraintes liées à l'agenda parlementaire et des avancées qu'il permet néanmoins, seul un vote conforme nous garantit que ce texte, ainsi que la proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Arcep, de notre collègue Patrick Chaize, soit adopté avant la fin du quinquennat. cette raison, comme l'ensemble de mes collègues, je voterai en l'état ces propositions de loi, préférant regarder le verre à moitié plein, c'est-à-dire l'apport réel de ce texte par rapport au droit existant, plutôt que le verre à moitié vide. La parole

la COP26 vient de s'ouvrir et nous venons de débattre de la nécessité d'un accord historique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour espérer contenir le réchauffement climatique et respecter l'accord ambitieux signé à Paris en 2015. Le dernier rapport du GIEC est venu une nouvelle fois tirer la sonnette d'alarme en suivant la trajectoire actuelle, nous en serons déjà à 2 degrés de plus en 2050, ce qui signifie la disparition totale des coraux, un rendement agricole qui s'effondre, 8 % de la population face à d'importantes pénuries d'eau et, pour être très concret, la fonte de presque tous les plus hauts sommets Face à ces données, des changements s'imposent à nous. Le numérique, qui permet bien sûr des progrès économiques, sociaux et écologiques, n'est pas en reste en matière d'empreinte carbone : on estime qu'il représente 2 % à 3 % des émissions de gaz à effet de serre en France- il pourrait même atteindre 7 % du total des émissions en 2040 si rien n'est fait. Pour bien comprendre, on peut se référer à la notion d'« empreinte cachée

L'Ademe a mis en lumière la face cachée écologique de plusieurs équipements de notre quotidien : pour un ordinateur de 2 kilos, il faut compter 600 kilos de minéraux, 200 kilos d'énergies fossiles et plusieurs milliers de litres d'eau douce d'un téléphone portable de moins de 300 grammes pèse au moins 70 kilos. C'est le sujet qui devrait nous préoccuper, puisque 81 % de l'empreinte environnementale du numérique repose sur le renouvellement des terminaux, notamment sur leur fabrication. L'Assemblée nationale a globalement conforté le travail du Sénat en juin dernier. Malheureusement, de nombreux reculs sont aussi à déplorer. Je pense notamment à la suppression du crédit d'impôt à la numérisation durable des durable des PME, à l'extension à cinq ans de la durée minimale de disponibilité des mises à jour de conformité, à la possibilité de rétablir les versions antérieures des logiciels pendant au moins deux ans, au rallongement de la durée légale de conformité. Toutes ces mesures visaient à freiner le renouvellement des terminaux. L'abaissement de l'ambition du texte par rapport à la version du Sénat doit-il pour autant nous pousser à rejeter ces propositions de loi ? Je ne le crois pas. Le calendrier législatif nous contraint à prendre une décision aujourd'hui : voter ces textes dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale pour les voir définitivement adoptés avant les prochaines échéances électorales et la suspension des travaux parlementaires. Aussi, malgré une certaine déception, le groupe du RDSE votera sans hésitation ces textes, qui participent incontestablement au verdissement du numérique, grâce au renforcement du délit d'obsolescence programmée- y compris logicielle au recours accru au recyclage, au réemploi et à la réparation des terminaux par les acteurs publics, au recours facilité aux pièces détachées pour les reconditionneurs ou encore à la mise en place d'opérations de collecte nationale s'accompagnant d'une prime au retour. J'aimerais profiter de cette tribune pour rappeler que, sur ce sujet, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Les élus locaux, notamment, s'engagent progressivement sur le chemin de la sobriété numérique.

fait aussi des efforts sur leur consommation d'énergie, qui n'a augmenté que de 1 % entre 2010 et 2018, alors que la quantité de calcul progressait de plus de 500 %. Aussi, avec l'adoption définitive de ces deux propositions de loi, et sans excès d'optimisme, nous pouvons croire en la réalisation de l'objectif que s'est fixé la France pour 2030 : zéro émission nette de gaz à effet de serre et 100 % de biens et services numériques écoconçus. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les transitions écologique et numérique convergent et s'inscrivent au coeur de nos sociétés et de nos politiques publiques.

Je crois au progrès, mais une innovation n'est pas bonne en soi ; elle doit faire sens. La responsabilité du politique est de ne pas rester à la surface des choses : elle est de résoudre les paradoxes de décider. Le numérique, la connexion d'acteurs en réseau, l'intelligence artificielle peuvent aider à optimiser des ressources limitées ; là est l'enjeu, en effet, mais nous ne saurions y répondre sans évaluer ni anticiper les effets du numérique, ainsi replacés dans une approche globale tenant compte des effets de substitution.

À cet égard, l'éducation des plus jeunes, dès l'école, à une utilisation responsable des outils numériques constitue en soi un projet de société. La prévention, ensuite, représente une innovation majeure pour nos politiques publiques. La plupart du temps, nous agissons en réaction, en correction.

Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), au travers duquel on ambitionnait de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois, a fait l'objet d'une loi, promulguée le 22 mai 2019, qui sera, demain, j'en suis certain, utilement complétée. L'entreprise participe historiquement à l'intérêt général, en étant moteur du progrès économique et technologique, créatrice de lien social et lieu d'accomplissement personnel.

Les entreprises, mais également les collectivités publiques, peuvent ainsi s'engager à réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est essentiel, la consommation électrique du numérique devant augmenter

à l'heure où les dirigeants du monde entier sont réunis dans le cadre de la COP26 pour travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, le Parlement poursuit son examen de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, dont nous débattons aujourd'hui en deuxième lecture.

Selon toutes les prévisions, cet impact environnemental va tendre à croître fortement au cours des années à venir, rendant plus que jamais nécessaire la mise en place d'une législation ambitieuse, traitant le problème sous tous ses aspects, de la consommation d'énergie à la valorisation des déchets. Dans le texte voté par le Palais Bourbon, nombre de dispositions importantes adoptées ici ont été conservées. Je pense notamment aux mesures de sensibilisation du public ou encore au renforcement de la répression de l'obsolescence programmée. Un ajout est à souligner : l'article 15 , qui renforce la lutte contre les appels frauduleux, source de nuisances de plus en plus importante pour nos concitoyens. En ce qui concerne les mesures relatives à la consommation d'énergie des centres de données,

En revanche, cela a été indiqué, les députés ont fait preuve d'une excessive timidité sur la question des appareils d'occasion, qui est pourtant- je l'avais souligné lors de la discussion du texte en première lecture -le nerf de la guerre. En particulier, alors que le Sénat s'était prononcé en faveur d'une exonération totale de la rémunération pour copie privée (RCP) pour les appareils d'occasion, l'Assemblée nationale est revenue sur cette exonération, remplacée par un taux spécifique, sauf pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Rappelons-le encore une fois, les terminaux numériques, c'est-à-dire les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones que nous avons dans nos poches, sont à l'origine de 81 % des émissions françaises du secteur.

Philippe Luce, président d'Institut Datacenter, « il n'y a pas de bâtiment qui, au mètre carré, coûte plus cher qu'un centre de données de haut niveau »,

je salue le travail accompli par notre commission et par nos rapporteurs sur ce texte, qui va permettre de réduire enfin concrètement les impacts environnementaux du secteur numérique. Au moment où la COP26 débute, sans grand espoir de parvenir à une stratégie mondiale pour limiter le réchauffement climatique, nous pouvons néanmoins, à l'échelon des États, agir concrètement et avec pragmatisme, secteur par secteur. À cet égard, le numérique fait partie des activités que l'on doit cibler pour réduire, d'une part, une empreinte considérable sur les matières premières et, d'autre part, un bilan carbone qui ne cesse de s'alourdir avec la multiplication des usages et des supports. J'ai un regret, toutefois, concernant la rémunération pour copie privée, qui, malgré l'opposition répétée du Sénat, frappera les produits issus du recyclage, alors qu'elle s'applique déjà aux produits neufs. Taxer des produits reconditionnés entre en contradiction avec les ambitions et les objectifs environnementaux de ce texte, mais, manifestement, les députés de la majorité et le Gouvernement ont préféré satisfaire des intérêts catégoriels, en l'occurrence ceux des acteurs culturels. Néanmoins, le texte prévoit un taux réduit de redevance pour l'ensemble de la filière et préserve le secteur de l'économie sociale et solidaire de cette pénalité ; c'est pour cette raison que j'ai retiré mon amendement de suppression En effet, il aurait été inadmissible que les emplois créés par les activités de reconditionnement dans les ateliers d'insertion professionnelle soient menacés, car, s'il existe une catégorie qui doit être soutenue, c'est bien celle des emplois permettant aux plus précaires de se réinsérer par le travail.

en tant que membre de la commission de la culture, je m'interroge sur l'utilisation de la rémunération pour copie numérique pour irriguer le secteur culturel.

au monde de la culture : elle lui aurait seulement retiré une recette hypothétique. Ensuite, l'article adopté par le Sénat ne conduisait pas à une exonération totale des équipements reconditionnés : auraient été exonérés les seuls biens ayant déjà fait l'objet d'un prélèvement lors de leur première mise en circulation. En d'autres termes, un prélèvement aurait été exigé pour les équipements reconditionnés en dehors des frontières européennes. Je note que cette solution intermédiaire a d'ailleurs été retenue par plusieurs pays européens.

à ce que nous ne nous opposions pas au principe de la RCP. Personne ne nie la nécessité de mieux subventionner la culture.

pour des raisons bien détaillées dans de nombreux articles de presse, notamment ceux, excellents, du journaliste Marc

Cet amendement vise à mettre en question le barème qui a été adopté. L'article 14 B entérine la décision de la Commission pour la rémunération de la copie privée assujettissant les produits reconditionnés à une redevance. Pour un smartphone de seconde main, celle-ci s'élèvera à 10,08 euros. Si la profession d'apothicaire a quasiment disparu, une forme d'expertise en matière de calculs au doigt mouillé semble avoir persisté au sein de la Commission pour la rémunération de la copie privée. Je vous conseille de lire le compte rendu de la réunion ayant entériné le taux qui nous est soumis aujourd'hui : c'est du grand art ! Retenez au moins qu'il a été fixé sans qu'aucun professionnel de la filière du reconditionné

À 10,08 euros, la redevance représente 6 % du prix final de revente, et ce alors que les marges du secteur oscillent entre 3 % et 6 %. Nous proposons donc de la fixer à 1 %.

Les industriels du secteur sont contraints par les lois du marché et par les comportements d'achat de proposer des produits reconditionnés à une faible fraction de leur prix de vente initial. Ces produits permettent donc d'alléger les charges pesant sur le pouvoir d'achat des Français, tout particulièrement des ménages les plus modestes.

devant le Conseil d'État. En votant cet article et en inscrivant ce barème dans le marbre de la loi, nous empêchons de fait les structures du reconditionné de faire valoir leurs droits devant la justice administrative. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa pour le remplacer par une mesure de gel de l'assujettissement à la RCP pour le secteur.

Cet amendement tend à préciser l'article 16, qui a pour objet de définir un « référentiel général d'écoconception des services numériques Toutefois, l'article, en l'état, n'indique pas la portée du dispositif visé. Il ne précise rien de ce que comportera ce référentiel. Il ne dit mot du cadre de conformité à la loi ni même d'éventuelles sanctions prévues en cas de non-respect du référentiel.

face à la numérisation de l'État. Nous savons combien il est difficile, pour les personnes en situation de handicap et les personnes les plus âgées, d'avoir recours aux services numériques. L'administration et les grandes entreprises doivent toutes tendre vers l'écoconception, qui rend possible l'accessibilité numérique. Enfin, cet amendement vise à définir un cadre cohérent de mise en oeuvre, d'un régime de sanctions préétabli par la commission. Plus le référentiel d'écoconception sera précis, mieux ses objectifs seront définis, plus il sera facile de le mettre en application. Nous ne devons pas laisser de place au flou. Quel

le prévoyait la proposition de loi initiale. Toutefois, après avoir entendu de nombreux acteurs, nous avions fait le choix, en première lecture, d'exclure ces personnes du champ du dispositif, afin d'en faciliter

du trafic provient de quinze fournisseurs seulement. Imposer un référentiel d'écoconception aux personnes publiques et aux personnes privées dotées d'une mission de service public aurait, dans ce cas,

ont élargi à l'ensemble des écoles d'ingénieurs, sans la réserver aux écoles d'ingénieurs du domaine de l'informatique, l'obligation d'une formation comportant un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.

Cet amendement avait été rejeté au motif qu'un cadre de régulation existe déjà. Celui-ci, néanmoins, n'est pas satisfaisant, ce dont le Gouvernement s'est récemment ému. En mai 2021, M. Jean Castex a déclaré : « La réalité est que, pour des millions de Français, souvent situés dans des territoires isolés,

dans nos territoires, le compte n'y est toujours pas. Certains habitants ne disposent même pas de l'accès de base à une ligne fixe. Je vous ai déjà saisi sans succès, monsieur le secrétaire d'État, du cas d'un monsieur de 82 ans habitant la commune de Cervon, dans la Nièvre, qui se voit refuser l'accès à une ligne fixe à son domicile et, par suite, l'accès à un service de téléalarme. Le présent article visant les engagements des opérateurs à réduire leurs émissions à effet de serre et leurs consommations énergétiques, je vous interpelle de nouveau à ce sujet. Je partage l'objectif d'un accès au numérique partout sur le territoire, avec une empreinte environnementale réduite. En zone rurale, de nombreux habitants ne sont toujours pas éligibles à la fibre et ne le seront pas avant quelques années. L'objectif de 2025 sera probablement difficile à tenir. Actuellement, en l'absence d'accès au très haut débit, l'usage de données mobiles telles que celles des réseaux 3G et 4G est favorisé par les opérateurs, car moins onéreux dans sa mise en oeuvre. Or cette utilisation de données mobiles a un impact environnemental plus important.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, je donne la parole à

est en fait bien intégré dans notre monde réel. J'émets donc le voeu que cette loi REEN puisse rester la reine des lois, et qu'elle trouve rapidement son roi ! La parole

Avant de passer au vote, je voudrais vraiment me féliciter de la qualité des débats en deuxième lecture sur cette proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize.